Messieurs les ministres, mes chers collègues, chers anciens collègues, cher président Bel – que je distingue dans notre tribune d’honneur c’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous avons appris, le 9 février dernier, la disparition de notre ancien collègue Robert Badinter. Robert Badinter fut un homme d’État au parcours exceptionnel. Il marqua de son empreinte non seulement notre assemblée, mais notre histoire tout entière. Chacun de nous sait ce que nous devons à cet homme à l’engagement sans faille. Robert Badinter vécut la justice avec exaltation. Quand il l’évoquait, il vibrait de toute son âme. Les Français retiendront ses brillantes plaidoiries, la force de ses discours à l’Assemblée nationale et ici, au Sénat. Robert Badinter connaissait la magie des mots, magie capable à elle seule de donner du souffle à son idéal républicain. Toute sa vie il s’en servit pour défendre les libertés publiques. Son combat le plus emblématique fut, bien entendu, celui en faveur de l’abolition de la peine de mort. En 2016, il avait souhaité remettre aux archives du Sénat l’exemplaire – que vous pouvez voir sur les écrans de l’hémicycle

Ce discours, qu’il nous a confié en dépôt, fut l’un des moments importants de l’histoire parlementaire française de la seconde moitié du XX siècle. En cela, ce fut un moment politique, au sens le plus noble du terme. Les Français restaient majoritairement attachés à la peine de mort en 1981. Elle avait été prononcée à huit reprises dans les années précédentes. Et pourtant, Robert Badinter savait que l’honneur du Parlement n’est pas le suivi systématique de l’opinion, mais au contraire qu’il devait l’éclairer. Un propos à méditer, pour aujourd’hui et demain… Il termina son discours dans notre hémicycle par ces mots : [S]i vous considérez, en conscience, qu’aucun homme n’est totalement coupable, qu’il ne faut pas désespérer de lui pour toujours, que notre justice, comme toute justice humaine, est nécessairement faillible et que tout le progrès de cette justice a été de dépasser la vengeance privée et la loi du talion, alors vous voterez pour l’abolition de la peine de mort. Plusieurs sénateurs exprimèrent au cours de ce débat une véritable émotion et des sentiments personnels, presque intimes. Robert Badinter déclara alors J’ai entendu des propos qui traduisaient souvent des convictions, parfois aussi des émotions respectables et même profondes. » Mais l’émotion réelle ne l’a pas emporté sur la réflexion et la détermination des votes. Et après trois jours de débat, c’est la responsabilité politique qui l’a emporté. Les sénateurs « ont eu pour conscience de voter en leur âme et conscience et ils ont aboli la peine de mort Celui qui fit abolir la peine de mort, après un discours inscrit à jamais dans les annales du Parlement, plaida dans les prétoires, des années durant, jusqu’à la limite – vous le savez – de ses forces. Il milita avec la même détermination aux côtés de François Mitterrand et de Pierre Mauroy. Il fut aussi celui qui dépénalisa l’homosexualité. Garde des sceaux exigeant, puis président du Conseil constitutionnel, il incarna une autorité morale et politique que nul n’a jamais songé à contester. Il fut un républicain exigeant, vouant, au delà de ses propres convictions, un respect sans faille à la loi, toujours attentif aux plus vulnérables. ans plus tard, Robert Badinter siégera dans cet hémicycle. Sénateur des Hauts de Seine, il fut un membre éminent du groupe socialiste et de la commission des lois. Chacune de ses interventions était écoutée avec respect. Avec Josselin de Rohan, Robert Badinter fut à l’origine de notre comité de déontologie parlementaire, qu’il me proposa à l’automne 2008. Il en fut d’ailleurs le premier président, de 2009 à 2011. Il a construit l’indépendance et l’impartialité de cet organe pluraliste, dans lequel tous les groupes politiques du Sénat sont représentés. Il s’attacha à dégager les grands principes déontologiques – indépendance, laïcité, assiduité, dignité, probité, intégrité – qui forment le socle de nos valeurs. En 2007, il fut naturellement désigné rapporteur du projet de loi constitutionnelle relatif à l’interdiction de la peine de mort. L’inscription, sur l’initiative du Président Jacques Chirac, de cette interdiction dans la Constitution ferma définitivement la porte à la peine capitale. Jusqu’à son dernier souffle, Robert Badinter continua sans relâche de se battre en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort avec la même conviction que dans l’hémicycle de notre Haute Assemblée. au cours d’une séance exceptionnelle consacrée ici même au trentième anniversaire du vote définitif par le Sénat du projet de loi portant abolition de la peine de mort, il déclarait ceci : « Ma conviction est absolue : comme la torture, dont elle est l’expression ultime, la peine de mort est vouée à disparaître de toutes les législations. Et les générations nouvelles verront un monde libéré de la peine de mort. » En relisant l’original de son discours de 1981, chacune, chacun d’entre vous, mes chers collègues, se verra transmettre cette force qui l’a animé. qui l’a animé. Vous pourrez ainsi reprendre le flambeau, le flambeau de l’humanisme et de la liberté. Conscient qu’il fallait dans certains cas aller au delà de la simple coopération traditionnelle entre États, il défendit au nom de la commission des lois des textes instaurant notamment des tribunaux universels. Il se prononça ainsi en faveur de la création d’un tribunal international en vue de juger les actes de génocide commis au Rwanda. Il plaida ensuite pour la création de la Cour pénale internationale, estimant qu’une juridiction permanente serait « un progrès considérable dans la lutte contre l’impunité des criminels contre l’humanité ». enfin, le rapporteur de la proposition de loi proposant d’édifier, dans la Clairière des fusillés au mont Valérien, un monument qui porterait le nom des résistants et des otages fusillés dans ces lieux

Robert Badinter souhaitait ce faisant que les jeunes générations puissent se souvenir qu’étaient ainsi morts des femmes et des hommes aux « convictions politiques, philosophiques, religieuses différentes, mais qui, tous, étaient unis dans le même amour de la France et de la liberté

Jusqu’au bout, il défendit les valeurs de la République, ces valeurs auxquelles sa grand mère Idiss était si attachée. Dans le beau livre qu’il lui a consacré, il évoque le sentiment de trahison ressenti par sa famille, par son père surtout, si fier d’être devenu citoyen français, citoyen de la patrie des droits de l’homme, après avoir fui les pogroms d’Europe orientale, père qui mourut, comme tant d’autres membres de sa famille, exterminé par la barbarie nazie, avec la complicité du régime de l’État français. Au fond, Robert Badinter restera sans doute cet éternel écorché vif qui aura gardé à jamais ses blessures d’enfant juif. Mais il restera cet infatigable combattant de la liberté Robert Badinter marquera à jamais notre assemblée et notre pays. J’ai le souvenir de son discours d’adieu, ici, en septembre 2011.

être le phare qui éclaire les voies de l’avenir, et non le miroir qui reflète les passions de l’opinion publique. » Voilà, après quinze j’exprime notre sympathie. À tous ceux qui l’ont connu, au delà de cet hémicycle, j’adresse mes pensées. À son épouse, Élisabeth Badinter, envers laquelle j’ai un immense respect et qui a rejoint notre marche le 12 novembre dernier, ici même au Sénat, à ses enfants, à toute sa famille et à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je souhaite redire la part que le Sénat prend à leur tristesse et à leur chagrin.

un juste, un ; rendre hommage à l’avocat au sens le plus noble du terme rendre hommage à l’homme des grandes causes humanistes, à l’homme de l’abolition de la peine de mort, à l’homme de l’abrogation du délit d’homosexualité, au défenseur du droit des victimes, à la conscience des conditions carcérales. rendre hommage au serviteur de l’État et au politique : au garde des sceaux qu’il a été, au président du Conseil constitutionnel et au sénateur qui a éclaboussé cet hémicycle de son talent oratoire. rendre hommage à l’intellectuel, à l’enseignant engagé pour les Lumières, au biographe de Condorcet. La France perd une conscience française l’un de ces hommes pour qui le progrès n’est pas un mot vain, puisqu’il en a été un artisan actif et inébranlable l’un de ces hommes qui ont parlé au cœur de la France, patrie des droits de l’homme, avec les mots et les valeurs qui nous rassemblent ; l’un de ces hommes qui ont donné à la politique ses lettres de noblesse, car la politique est toujours noble quand elle défend la justice et quand elle fait avancer les causes humanistes. Une conscience française, enfin, car Robert Badinter n’hésitait pas à nous mettre face à nos démons, à nos bassesses, à nos renoncements collectifs, passés et présents. C’était une vigie de la justice. On se souvient de son fameux : « Vous m’avez fait honte ! » À cet avertissement du grand homme, à ce rappel que le pire dans l’Histoire est toujours possible, la France ne peut que répondre : « Monsieur Badinter, vous nous avez rendus fiers.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, les projets de loi ordinaire et de loi organique proposent trois réformes techniques, destinées à accompagner la relance de la filière française du nucléaire, actée par la loi du 22 juin 2023 La première réforme est la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) au sein d’une même autorité, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection La suivante est la simplification des règles de la commande publique pour les projets nucléaires. La dernière est le repositionnement du haut commissaire à l’énergie atomique (HCEA). Ce texte a mobilisé la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, saisie au fond de la première réforme, et la commission des affaires économiques, saisie pour avis de la première réforme et au fond des deux autres. autres. Je remercie MM. les présidents de commission et M. le rapporteur Pascal Martin. Lors de l’examen de la loi Nouveau nucléaire, le Gouvernement avait déposé à l’Assemblée nationale deux amendements visant à fusionner l’ASN et l’IRSN. En commission mixte paritaire, le rapporteur de la commission des affaires économiques avait expurgé le texte de toute référence à la fusion. De plus, sa présidente avait saisi l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques En rejetant les amendements présentés à la hâte par le Gouvernement, le Sénat, par un vote massif, avait refusé une réforme mal anticipée et mal évaluée. En saisissant l’Opecst, nous avions remis les parlementaires au cœur des enjeux. Pour ce nouveau projet de réforme, le Gouvernement n’a pas vraiment changé de méthode : il a affiché un souverain mépris pour la représentation nationale. Entre la désignation du nouveau Premier ministre, le 8 janvier dernier, et l’examen du texte, mercredi dernier, il s’est écoulé un mois… Un mois de vacance du pouvoir ! En effet, nous n’avions ni ministre identifié ni direction compétente. Le Gouvernement a refusé d’être auditionné, à rebours de tous les usages. L’absence de cabinet a empêché des échanges en amont et des retours dans les temps cela a nui à nos travaux préalables et, plus généralement, à la clarté et à la sincérité des débats. Or le sujet sur lequel nous légiférons est bien trop sérieux pour une telle improvisation. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la semaine passée la simplification normative. Nous partageons tous ici cet objectif. Cependant, simplifier les normes ne signifie pas enjamber le Parlement. Les amendements parlementaires, sénatoriaux, ne sont pas un obstacle à la mécanique bien huilée de vos projets de réforme. Ils sont au contraire un gage d’exigence juridique, d’expérience politique et d’acceptabilité sociale. avons tout à gagner à accepter la délibération, à se frotter à la contradiction, à rechercher le compromis. Sur le fond, cependant, le nouveau projet de réforme est plus abouti que le précédent il est le fruit du rapport de l’Opecst, d’une dizaine de consultations et d’un an de concertations. Il arrive au moment crucial de la relance du nucléaire, le Gouvernement devant proposer de nouvelles régulation et programmation énergétiques, dans un projet de loi sur l’énergie et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Nous soutenons aujourd’hui, dans son principe, le nouveau projet de réforme. Parce qu’il vise à fluidifier les procédures d’instruction, à sûreté inchangée, il est indispensable à la relance du nucléaire. Certes, les modalités du projet posent des défis, en matière de continuité des procédures, de valorisation des compétences et de maintien des standards. Pour autant, à terme, le projet est de nature à renforcer la confiance du public, car la nouvelle autorité sera une autorité administrative indépendante (AAI). Dans le cadre de mes travaux, en tant que rapporteur de la commission des affaires économiques, j’ai entendu une quarantaine de personnalités, lors d’une vingtaine d’auditions.

amendements ont été adoptés en commission et six en séance publique. Le premier axe de mes travaux vise à consolider la gouvernance de la filière du nucléaire, en renforçant les attributions et le fonctionnement du haut commissaire et en prévoyant que le Parlement puisse le saisir pour avis et se prononcer sur sa désignation. Le recours à la procédure de l’article 13 de la Constitution n’a d’ailleurs rien d’inédit. Je sais, monsieur le ministre, que cela vous a agacé.

ans après sa création par le général de Gaulle, l’objectif est de faire du HCEA la vigie de la relance du nucléaire. Le deuxième axe tend à simplifier les règles de la commande publique des projets nucléaires, en confortant les dérogations prévues en matière d’allotissement, de durée des accords cadres et de règles de publicité et de concurrence, et en ajoutant un critère de crédibilité et une possibilité d’avenant. Ces souplesses sont nécessaires pour prévenir tout risque d’interface, de rupture et,, de surcoût.

en proposant d’appliquer les recommandations du rapport de l’Opecst et de réintroduire des dispositions visant à appliquer une règle de parité dans le collège de l’autorité et une règle de publicité dans sa commission des sanctions. Voilà un gage de cohérence. au dernier axe, nous proposons de conforter l’organisation de l’autorité de sûreté, notamment en matière de garantie d’indépendance et de déontologie, de séparation entre les processus d’expertise et de contrôle, de publication des rapports et des décisions ou d’association de l’Opecst et des commissions parlementaires Nous avons aussi consacré l’indépendance de l’autorité, en complétant son intitulé, et sanctuarisé ses activités régaliennes, en prohibant le recours, pour ces dernières, aux personnels étrangers. conclure, le projet de réforme, tel qu’amendé, mérite d’être soutenu ; je vous invite donc à l’adopter. Quoi qu’il en soit, monsieur le ministre, le Gouvernement devra, dans d’autres véhicules législatifs et dans d’autres débats, concrétiser enfin la relance du nucléaire.

ce projet de fusion entre l’ASN et l’IRSN arrive à son terme, avec bien du retard, cet après midi. Il y a une quinzaine d’années, le Président Sarkozy avait envisagé cette réforme, mais l’incident de Fukushima l’avait fait reculer, sur ce sujet comme sur tant d’autres. Il faut dire que l’IRSN s’était peu à peu transformé en jouant les Cassandre de l’apocalypse nucléaire, diffusant ici et là parmi le public des informations alarmistes, instillant le doute dans la population, outrepassant bien souvent ses prérogatives, par excès de sûreté voire de militantisme. pouvons par exemple évoquer le rôle de l’institut dans l’étude sur l’efficacité de la station de surveillance des rejets de la centrale de Chinon, après qu’il avait été interpellé par une association antinucléaire en 2019 – cette étude aura duré deux longues années et coûté 650 000 euros ou bien son rôle dans l’arrêt de quatre réacteurs de la centrale du Tricastin en 2017 ; ou encore dans le retard considérable pris sur le chantier de l’EPR de Flamanville en 2018. Ce, chaque fois, pour des motifs fortement contestés par les autres acteurs de la filière nucléaire. Tous ces épisodes ont généré des pertes de dizaines de millions d’euros. le plus dommageable intervient en 2021, quand l’IRSN oblige EDF à fermer un grand nombre de réacteurs à cause de corrosions découvertes sur des circuits, alors que l’opérateur propose de faire les contrôles tout en continuant la production d’électricité. Cette obstination de l’IRSN aura pour conséquence directe la perte de plus de 30 milliards d’euros et un renchérissement considérable de notre facture d’électricité au moment où éclate la guerre en Ukraine, dont nous subissons encore les conséquences. La majorité présidentielle n’est évidemment pas en reste dans cette succession de mauvaises décisions, elle qui aura commencé en 2017 en fermant Fessenheim, alors que tous les spécialistes affirmaient que cette centrale pouvait fonctionner encore pendant des années, cédant là aussi à un principe de précaution excessif, pour de basses considérations électoralistes. Sept ans plus tard, cette même majorité présidentielle a une fois de plus retourné sa veste et est devenue pronucléaire, redécouvrant subitement l’un des seuls avantages comparatifs industriels de notre pays.

Pourtant, les défis ne manquent pas pour redonner à la France sa place de leader dans le nucléaire, afin d’avoir une énergie décarbonée, pilotable et sûre, tels que la construction de nouveaux réacteurs à eau pressurisée, les EPR2, le développement de petits réacteurs modulaires, les SMR, à sels fondus, au sodium, ou le soutien à différents programmes de recherche comme Jules Horowitz ou Iter, avec en ligne de mire la maîtrise de la fusion d’ici à la fin du siècle, énergie propre et quasi infinie, qui permettra de mettre définitivement au placard tous les décroissants antisciences de notre époque. Nous voterons donc pour ce projet de loi, mais en espérant que la Macronie ne se reniera pas dans six mois et conservera ce cap pronucléaire dont notre pays a besoin. La parole

Cette vision équilibrée doit maintenant s’accompagner d’actes. Si le Président de la République nous a donné la direction, nous devons désormais élaborer un plan clair de navigation. Depuis février 2022, les lois votées ont contribué à en former l’architecture et les contours. La prochaine étape est attendue rapidement et avec un intérêt tout particulier par la Chambre haute. Le projet de loi Souveraineté énergétique permettra à toute la structure de tenir pour les prochaines années. Il ne faut pas se le cacher, cela représente un véritable effort financier pour notre pays sur des dizaines d’années à venir. Il nous faut développer des technologies nouvelles, tout en maintenant nos installations existantes le plus longtemps possible et dans la sécurité. Ce dernier point est d’ailleurs particulièrement remis en question par le changement climatique, le manque d’eau ou encore les canicules. Tous ces défis ne peuvent donc se passer de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, qui font partie intégrante de la relance. La déclinaison de ce programme ne doit pas nous faire oublier un point essentiel, à savoir l’approbation des populations. Pour que les habitants continuent à accepter la présence du nucléaire sur leur territoire, ils ont besoin d’être rassurés en termes de sécurité et de sûreté.

Travailler à la gouvernance de cette sûreté fait donc partie des fondations de la relance du nucléaire, et ce projet de loi y contribue. Je salue, à ce titre, l’engagement du Gouvernement, les travaux menés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi que nos débats en commission et en séance publique. La nouvelle entité de sûreté nucléaire et de radioprotection aura une tâche immense face à elle. Avant d’envoyer ce texte devant l’Assemblée nationale, nous pouvons déjà relever des points de satisfaction. Le premier volet que j’aborderai ici est le règlement intérieur. Les garanties qui sont désormais présentes dans le texte dessinent un cadre. Nous y sommes et y serons attentifs, tant il y va de la réussite de la fusion des deux entités. Le recours à des groupes permanents d’experts et la mise en place d’une commission d’éthique et de déontologie sont des éléments positifs.

» Organiser une fusion, c’est d’abord réunir dans une nouvelle entité des professionnels qui, parfois, n’ont ni la même culture, ni la même histoire, ni la même approche du travail. Si la stratégie développée ici est d’aller vite pour gagner en efficacité, il faut toutefois faire attention à ce que l’urgence du projet n’entraîne pas des difficultés pour les personnels en place. Ils jouent un rôle essentiel dans la stratégie nucléaire et dans la stratégie énergétique de notre pays. S’ils ne se retrouvent pas dans la nouvelle entité, la fusion échouera et nous perdrons du temps, de l’argent et des compétences. Je le répète, les personnels des deux entités doivent donc trouver leurs places, afin de rester engagés, fidèles et professionnels, comme ils l’étaient dans leurs instances initiales. Nous devrons également faire attention à l’attractivité des professions de la future agence. Comme le disait mon collègue Pierre Jean Rochette lors de la discussion générale, nous avons la chance de former des profils d’excellence. Ce sont eux qui font la force de notre nucléaire français. Tout l’enjeu Tout l’enjeu est qu’ils veuillent bien demeurer chez nous afin de mettre leur cerveau au service de la France. C’est grandiloquent, je vous l’accorde, mais,, c’est la souveraineté de notre pays qui est en jeu.

Parler de transparence dans la sûreté, c’est surtout en faire une réalité, afin que les Français adhèrent à la relance du nucléaire. Selon moi, la nouvelle agence sera un exemple du genre. La France est déjà un leader mondial dans ce domaine, et doit le rester. Rendre publics des rapports d’activité et permettre aux institutions d’y avoir accès est une bonne chose. Le fonctionnement externe comprend aussi un lien privilégié avec la filière du nucléaire, afin de connaître les innovations, développer la recherche et s’assurer de l’effectivité des dispositifs de sûreté et de radioprotection. Cependant,

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, voilà quelques semaines, à l’amorce de l’examen du projet de loi et du projet de loi organique, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’était fixé une priorité essentielle maintenir notre sûreté nucléaire au niveau d’exigence le plus élevé possible, en l’adaptant aux enjeux de notre décennie et de celles à venir. L’excellence de notre système de sûreté nucléaire est reconnue par tous. vous le savez, il fait face à une charge sans précédent. Dans les années 1970, le plan Messmer avait conduit à la construction d’un parc nucléaire en quelques années. Aujourd’hui, le défi est tout autre : la sûreté nucléaire devra à la fois s’adapter au chantier inédit du programme nucléaire gouvernemental, poursuivre l’exploitation du parc nucléaire existant et prévenir les risques liés au changement climatique. Face à ce flux de demandes, une réforme était nécessaire. Tout en garantissant un niveau d’exigence le plus élevé possible, la réforme de la gouvernance de la sûreté devra renforcer l’efficacité des procédures, s’adapter à l’évolution des acteurs du nucléaire, avec l’essor des start up, améliorer la réponse en cas de crise, clarifier la communication auprès du public et, enfin, renforcer l’attractivité des métiers de la sûreté. Le texte initial du Gouvernement permettait il d’atteindre l’objectif que notre commission s’était fixé, à savoir le maintien de notre sûreté nucléaire au niveau d’exigence le plus élevé possible, en l’adaptant aux enjeux de notre décennie et de celles à venir ? J’ai donc proposé, en tant que rapporteur de ce texte, des ajustements au projet du Gouvernement pour parvenir à un équilibre, qui me semble aujourd’hui satisfait, par une approche à charge et à décharge. Je nourris un regret majeur, celui de n’avoir pu auditionner en commission le ministre chargé de ce dossier. Première amélioration notable : la distinction entre expertise et décision. Le projet de loi introduisait, dans sa rédaction initiale, un recul, d’abord sur la méthode, en renvoyant le sujet au règlement intérieur de la future autorité, et surtout sur le fond, en prévoyant une distinction des « processus » d’expertise et de décision uniquement dans le cas d’une prise de décision par le collège, soit trente dossiers par an, contre trois cents Un redémarrage de centrale nucléaire n’aurait ainsi plus fait l’objet d’une expertise distincte du reste de l’instruction ! La version que nous nous apprêtons du moins l’espèré je à adopter préservera la fluidité permise par la fusion des deux entités, l’ASN et l’IRSN, tout en garantissant la confrontation des doutes, indispensable à la sûreté. Notre texte étend tout d’abord le champ de la distinction entre expertise et décision à l’ensemble des dossiers à enjeux, et non pas seulement aux trente sujets annuels nécessitant une décision du collège. Nous nous sommes également assurés que le signataire de l’expertise ne sera pas le signataire de la décision. Par ailleurs, nous avons garanti, sur un dossier donné, que les personnels chargés de l’expertise, d’une part, et ceux qui seront chargés de la décision, d’autre part, soient bien identifiés, sans pour autant recréer au sein de la nouvelle autorité un pôle « expertise » distinct d’un pôle « décision ». Enfin, nous avons renforcé l’expertise tierce, en donnant une assise juridique forte aux groupes permanents d’experts, les GPE, comme le proposait le rapport de l’Opecst. Deuxième amélioration essentielle : le maintien d’un niveau exigeant de transparence. En renvoyant au règlement intérieur les modalités de publication des résultats des activités d’expertise de la nouvelle autorité, le projet de loi initial comportait des risques de recul en la matière, puisqu’il n’était pas certain que l’exigence de publication soit conservée, et encore moins qu’elle soit renforcée. Comme le proposait le rapport de l’Opecst, nous avons donc inscrit dans la loi un principe de publication des résultats d’expertise. Troisième amélioration nous avons contribué au maintien des activités de recherche au sein de la nouvelle autorité. Le projet de loi initial comportait des risques pour la conduite de ces activités, qui sont le socle de l’expertise en matière de sûreté et de radioprotection. Nous avons fort heureusement adopté plusieurs amendements visant à prévenir les conflits d’intérêts, en permettant au président de l’autorité de donner délégation de pouvoir aux services pour la signature de conventions,

Le quatrième risque induit par le texte initial était relatif à l’association du Parlement et de la société civile. Nous avons, là aussi, redressé le projet de loi, en prévoyant d’associer à l’élaboration du règlement intérieur l’Opecst, le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), l’Association nationale des commissions et comités locaux d’informations (Anccli), et les commissions permanentes compétentes des deux assemblées. Enfin, avec ce texte, nous améliorons sensiblement la gestion de crise et apportons une clarification indispensable dans le domaine de la communication.

La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

11 mars 2011 et de son horreur absolue. Le Japon est alors frappé par un séisme et un tsunami dévastateur, qui provoquent une catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima.

154 000, nombre de personnes évacuées de la zone entourant la centrale nucléaire ; des centaines de milliards de dollars, coût estimé de la catastrophe.

La sûreté nucléaire est une affaire sérieuse. En France, nous avons la chance extraordinaire de disposer de 1750 femmes et hommes ayant pour mission l’expertise, la recherche, la protection, l’anticipation et le partage d’informations au service des pouvoirs publics et de la population. Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial singulier et d’une exception à la française. une méthode à la française – je reviendrai sur ce point –, qui repose sur une sûreté nucléaire adaptative et non normative, sur un système dual préservant l’expertise de la décision. Sa singularité réside dans la collaboration entre chercheurs et experts, pour anticiper les évolutions et maîtriser les risques nucléaires et radiologiques.

compromettre notre sûreté et la sécurité des Françaises et des Français. Vous accélérez, mais le débat parlementaire est entravé. L’examen de ce texte n’a pas bénéficié du temps nécessaire, aucun ministre n’a été auditionné en commission,

pense notamment au calendrier serré dans lequel vous vous inscrivez. Qui peut imaginer une mise en œuvre sérieuse et sûre au 1 janvier 2025 ? En à peine dix mois, vous voulez fusionner deux organisations primordiales pour la sûreté nucléaire. Ce n’est pas sérieux, monsieur le ministre ! Vous voulez tout attaquer en même temps. Votre relance du nucléaire est risquée.

Vous l’aurez compris, nous sommes profondément opposés à ce texte, qui est dangereux. Toutefois, la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ont

Comme l’a dit Daniel Salmon, nous resterons attentifs au cours de la navette parlementaire, pour éviter tout recul, notamment sur le sujet primordial la séparation des compétences entre expertise et prise de décision, sur l’obligation de publication des résultats d’expertise avant les décisions, sur le maintien des partenariats de recherche entre l’ASNR et les acteurs industriels du secteur, et, enfin, sur l’information du Parlement et des citoyens, qui est le fondement même de la confiance des citoyens envers la sûreté nucléaire. Vous avez systématiquement renvoyé des dispositions importantes au règlement intérieur. Nous n’approuvons pas ces renvois, qui excluent de fait les parlementaires et la société civile. Mais vous n’écoutez pas, nous le savons bien. L’Opecst, comme de nombreux organismes consultés, a averti que la transition vers une nouvelle organisation pourrait « poser des difficultés ». Mais vous n’écoutez pas peu importe ce que vous disent les experts, vous imposez, sans écouter. Au détriment de la sûreté nucléaire, la recherche est mise sous tutelle, les corps intermédiaires sont muselés, les associations, les syndicats, les organisations non gouvernementales (ONG), les élus locaux et même, parfois, le Parlement, sont piétinés.

ont dénoncé la « mise au placard » de leur travail, alors que la santé des populations est en jeu. Vous faites le contraire de ce qui est préconisé par les scientifiques. Certes, vous l’assumez, mais c’est irresponsable. Monsieur le ministre, oui, nous sommes contre le nucléaire, mais nous sommes pour la sûreté nucléaire. Écoutez toutes celles et ceux qui vous alertent. La relance nucléaire est une impasse financière et les risques associés demandent de la démocratie et du temps. La souveraineté énergétique que vous appelez de vos vœux est un leurre ! Je le rappelle, la dernière mine française d’uranium a fermé ses portes en mai 2001. J’ai commencé par vous rappeler la catastrophe de Fukushima, parce que toutes vos décisions, toutes nos décisions, devraient être construites autour de la maîtrise du risque d’accident nucléaire. notre opposition à ce texte persiste. Malgré les efforts faits pour atténuer certains risques, nous vous invitons à refuser la fin de notre modèle d’expertise… et de contrôle et à ne pas voter en faveur de ce projet de loi aussi inachevé que dangereux. La parole

la relance et le développement de la filière nucléaire ne pourront se faire que dans la plus grande transparence et avec la confiance de nos concitoyens. L’efficacité et la crédibilité du système de contrôle de la sûreté nucléaire sont une condition indispensable à l’emploi de cette énergie. C’est une obligation morale, mais aussi légale. la Charte de l’environnement et les conventions internationales dont nous sommes parties prenantes nous obligent. Or, malgré des débats riches et de qualité, les oppositions à ce projet de loi sont renforcées et les doutes légitimes quant au bien fondé de la fusion entre l’ASN et l’IRSN subsistent. En effet, nous ne savons toujours pas pourquoi le Gouvernement veut remettre en cause un système de sûreté qui fonctionne et a fait ses preuves. L’IRSN mène des expertises en sûreté nucléaire et éclaire l’ASN, qui, de son côté, prend des décisions administratives.

qu’il n’y ait pas eu d’analyse complète des forces et faiblesses de l’organisation actuelle avant toute modification et fusion. Ce point constitue également un élément central de l’avis du comité d’éthique et de déontologie de l’IRSN, pour qui les objectifs de cette réorganisation restent, pour une large part, peu explicites. Nous ne savons toujours pas pourquoi le Gouvernement prend le risque de déstabiliser profondément la gouvernance de la sûreté nucléaire, à l’heure où les chantiers sont énormes poursuite de l’exploitation des réacteurs au delà de quarante ans, voire soixante ans, construction de nouveaux réacteurs, d’installations d’entreposage du combustible et de stockage géologique. Je pense également à l’apparition de nouveaux acteurs privés, qui engagent la conception de petits réacteurs, les SMR, dans le cadre du programme France 2030. Nous ne savons toujours pas quel sera le sort fait aux salariés de l’IRSN et aux fonctionnaires de l’ASN. Nos amendements sur ces sujets – l’un d’eux prévoyait le maintien d’une proportion de fonctionnaires au moins égale à l’existant dans la nouvelle autorité – ont été déclarés irrecevables ou balayés d’un revers de la main. Pourtant, la question est cruciale pour le maintien d’une culture administrative indispensable à l’exercice des missions régaliennes et des pouvoirs de police en matière de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. S’agissant des salariés de l’IRSN, ce projet de loi entraîne une hémorragie de départs. Le Gouvernement n’a été capable ni d’instaurer un véritable dialogue avec les personnels ni de faire preuve d’une certaine clarté sur ses motivations.

sous tension. En revanche, nous savons que l’indépendance de l’expertise n’est pas assurée et que le renvoi au règlement intérieur n’est pas satisfaisant. Vous avez refusé de préciser, comme nous vous invitions à le faire, que l’expertise ne sera pas soumise au dogme de la faisabilité industrielle et du bilan coût/avantage, tout comme vous refusez la mise en place d’un pilotage de la recherche, au travers d’un conseil scientifique et d’un comité d’orientation des recherches avec de nombreuses parties prenantes. Nous savons également que la transparence n’est pas assurée. À cet égard ; comme le soulignent de nombreux avis, « la loi fait très peu de cas de la société civile », alors que, à l’aune d’une relance du nucléaire, il est temps de lui donner une place et de lui montrer qu’elle est considérée comme « partie prenante » de cette relance historique. Or vous avez refusé de conforter le principe de publication des avis en amont de la décision, tout comme vous avez refusé la mention explicite de la charte d’ouverture à la société, que l’IRSN partage avec de nombreux organismes, dont l’Agence (BRGM), l’Inrae et Santé publique France, piliers du dialogue avec la société civile. Nous savons aussi que le Gouvernement et la majorité sénatoriale ont refusé la prise en compte explicite des travailleurs sous traitants, ces nomades du nucléaire, surexposés aux risques et au phénomène de « gestion de l’emploi par la dose ». Tout en reconnaissant leur caractère indispensable et leur exposition, vous refusez de les nommer. Or les nommer, c’est les reconnaître ! Enfin, le fait de séparer les expertises de sûreté des installations civiles de celles de défense présente le risque de voir diverger les approches de sûreté entre ces installations. La transparence et la politique d’ouverture à la société sont des acquis institutionnels incontestables, fruits d’un long travail des acteurs de la sûreté nucléaire. La réforme pourrait les remettre en cause sans justification pertinente. La sûreté nucléaire, c’est un contrat de confiance entre la société tout entière, les exploitants et les instances de contrôle. L’ASN et l’IRSN renforcent ce contrat de confiance, du fait même de la séparation claire de leurs rôles respectifs : d’une part, l’analyse scientifique des risques l’exercice de la prise de décision. Vous prenez le risque, monsieur le ministre, de rompre ce contrat. C’est sans doute d’une véritable autorité publique indépendante que nous aurions eu besoin, une autorité qui veille à protéger les droits des citoyens sans être soumise à l’autorité de l’État, ce qui lui permettrait d’exercer ses missions de manière impartiale et libre de tout conflit d’intérêts. Or vous étiez réticent au simple ajout du mot « indépendance » pour désigner la future ARSN ! Vous l’aurez compris, mes chers collègues, ce texte est à rebours de notre exigence d’une gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au service de l’intérêt général et non pas du seul volet

nos engagements de développement durable, mais aussi, car il convient d’être pragmatique, la vie quotidienne de nos administrés. Comme vous le savez, le groupe RDSE apprécie, plus que tout, le débat, ainsi que les propos nuancés, et ce d’autant plus quand ils concernent le nucléaire. Le débat qui nous anime aujourd’hui n’est d’ailleurs pas d’être pour ou contre la relance de notre filière nucléaire. Je le rappelle, le Sénat s’est déjà positionné sur ce point en votant en mai dernier, avec une large majorité, la loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. Il s’agit bien ici de la réforme de notre système de sûreté nucléaire. Ce système, dans sa configuration actuelle, duale, a acquis une reconnaissance nationale et internationale. Il agit en toute indépendance, transparence et impartialité, au service de l’intérêt général, et bénéficie de la confiance de nos concitoyens, pierre angulaire de l’acceptabilité sociale du nucléaire. Cette transparence n’était pourtant pas tout à fait au rendez vous quand, il y a tout juste un an, il a été proposé au sein du conseil de politique nucléaire, puis glissé dans un amendement à l’Assemblée nationale, de faire adopter cette réforme. Je suis heureux que le Parlement ait pu ainsi reprendre sa place, au côté de l’exécutif. Car, si la relance historique de notre filière nucléaire exige de nous que nous repensions et adaptions l’organisation de notre sûreté nucléaire, les débats qu’elle suscite sont essentiels puisque, rappelons le, faire la démonstration de la sûreté d’un système, c’est aussi le confronter au doute. Nous comprenons l’ambition, l’intention, la volonté portées par cette réforme, dans un contexte où le nombre de dossiers à traiter sera appelé à croître de façon inédite. Néanmoins, je dois avouer que j’ai eu bien du mal, et beaucoup de mes collègues avec moi, à me forger une conviction solide quant à la pertinence du projet de loi qui nous est soumis. soumis. Force est de reconnaître que beaucoup de questions demeurent, après analyse du texte, malgré le travail exigeant en commission ; le débat n’est sans doute pas clos, notamment sur le plan budgétaire. Je souhaite vivement que nous gardions en tête l’objectif de ne pas ébranler un système qui, par sa dualité et sa fiabilité, a tissé un véritable lien de confiance avec les Français, condition pour que cette relance historique de la filière se fasse de manière optimale. À ce titre, il faut louer les travaux effectués par le Sénat, qui s’est efforcé d’ériger les garde fous nécessaires au manque de transparence, en mettant en place les conditions d’une séparation nécessaire entre experts et décideurs. C’est un apport législatif majeur dont je salue la pertinence. Nous avons atteint aujourd’hui une position d’équilibre, préservant la fluidité, l’optimisation et l’efficience des processus décisionnels – c’était l’objectif de cette fusion –, tout en garantissant la confrontation des doutes indispensables à la sûreté. Toutefois, comme l’a rappelé mon collègue Raphaël Daubet lors de la discussion générale, le risque perdure, malgré l’engagement sincère des sénateurs, sénateurs, de créer tout simplement un nouveau système bicéphale au sein d’une entité fusionnée, recréant ainsi les risques de paralysie que cette réforme voulait outrepasser. À rechercher un équilibre parfait entre, d’une part, l’amélioration de l’efficience des procédures et, d’autre part, le maintien de notre sûreté nucléaire au niveau d’exigence et de transparence le plus élevé possible, cette fusion prend le risque d’entraîner une désorganisation du fonctionnement de deux organismes qui ont appris au fil des années à travailler en bonne intelligence. Il existe, nous le savons, quelques alternatives à la nécessité de refonte de la gouvernance de notre sûreté nucléaire. Je pense ici à une augmentation substantielle des ressources de l’IRSN et de l’ASN pour garantir leur soutenabilité sur le long terme, à la poursuite de l’effort d’augmentation des moyens humains pour ces deux entités, tout en revoyant leurs politiques de ressources humaines afin de renforcer l’attractivité de leurs métiers. Sans doute pouvons nous aller plus loin, notamment par un engagement budgétaire constant. Nous y serons attentifs.

du problème de sous traitance de la part des exploitants, qui engage la problématique de la sûreté nucléaire dans sa globalité L’ASN s’est déjà fendue d’un rapport très critique vis à vis d’EDF dans lequel elle a estimé que l’électricien public ne fait pas respecter les standards de construction de « haute qualité » par ses sous traitants. Nous entendons bien les partisans de la simplification et de l’efficacité ; leurs remarques, dans un contexte exceptionnel, ont du sens. Toutefois la mise en place d’une nouvelle architecture plus incertaine du contrôle de la sûreté nucléaire ne doit pas entraîner un bouleversement synonyme de perte de confiance de nos concitoyens. Mes chers collègues, il ne s’agit pas ici de réduire le nombre de normes applicables aux haies, mais il s’agit bien de sûreté nucléaire. Si nous nous rejoignons pleinement quant à la nécessaire évolution de notre système, nous n’avons toutefois pas l’assurance que la réponse apportée par la fusion soit la plus appropriée, qui plus est dans ce contexte d’urgence, avec la perspective d’un prochain EPR en 2035, alors que le travail administratif d’intégration peut perdurer quelques années. Le nucléaire a un rôle clé à jouer dans notre politique énergétique, au même titre que la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Or notre mix énergétique doit répondre aux exigences d’une énergie décarbonée, pilotable, disponible et sûre. Si le RDSE, vigilant, verra ses votes s’exprimer de manière hétérogène, assuré, monsieur le ministre, qu’ils seront sous tendus par la volonté commune d’une sûreté nucléaire renforcée, indépendante et transparente, et ce quelle qu’en soit son organisation, en vue d’affronter ce contexte hors norme lié à la relance de notre filière nucléaire. La parole

faire de la France le premier grand pays industriel au monde à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles alors que ces dernières représentent encore près de deux tiers de notre consommation d’énergie finale Pour relever ce défi, nous n’avons pas le choix : il nous faudra accélérer massivement la production d’énergies décarbonées, nucléaires comme renouvelables. C’est tout le sens des deux lois d’accélération sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire que nous avons votées l’année dernière. C’est tout le sens aussi de la réforme du marché européen de l’électricité, qui permet de mettre ces énergies décarbonées, dont le nucléaire, au cœur des politiques européennes. Je salue d’ailleurs le travail d’Agnès Pannier Runacher sur ces sujets. Au Sénat, nous n’avons pas le nucléaire honteux. La création d’une délégation de programme interministérielle au nouveau nucléaire, les crédits d’investissement massifs des plans France Relance et France 2030 en faveur du nucléaire et la tenue de conseils de politique nucléaire sont des signaux très positifs pour notre filière. Mais cette relance du nucléaire doit nous permettre de répondre à plusieurs enjeux : réduire nos émissions grâce à la production d’une énergie décarbonée ; baisser la facture pour les ménages ; tenir nos engagements de sortie des énergies fossiles participer à la réindustrialisation de la France puisque les chantiers EPR2 seront en effet les plus importants d’Europe ; renforcer la souveraineté énergétique de notre pays dans un contexte géopolitique de plus en plus instable. Une France souveraine face aux instabilités géopolitiques est une France qui maîtrise sa production. Si l’histoire du nucléaire a été un véritable succès, bénéficiant d’un large niveau de confiance, c’est avant tout grâce au cadre de sûreté mis en place, un cadre de sûreté qui repose d’abord sur la responsabilité des exploitants ainsi que sur une organisation permettant un contrôle indépendant. Toutefois, comme l’ont souligné de nombreux collègues lors de l’examen du texte, le contexte que nous avons devant nous est complètement hors norme, en termes tant de volumes que de complexité. Durant les prochaines années et les prochaines décennies, nous devrons faire face à plusieurs défis : la prolongation du parc existant ; le développement du nouveau nucléaire français avec les EPR2 et les SMR ; la construction de nouvelles solutions de stockage des déchets. Alors que nous n’avons lancé qu’un chantier d’EPR2 en France depuis vingt ans, c’est un changement de paradigme complet qui requiert un niveau de sûreté optimal et inchangé pour être réussi et accepté par nos concitoyens. Il s’agit aussi d’un enjeu industriel clé, avec 100 000 emplois à créer en dix ans.

Ce projet de loi fait suite à un premier débat qui s’est tenu en début d’année dernière lors de l’examen du texte d’accélération du nucléaire, sur la base d’un amendement gouvernemental qui n’avait malheureusement pas été présenté au Sénat. Le groupe RDPI se félicite qu’une réflexion de plus long terme sur un enjeu aussi important ait pu avoir lieu avec un rapport parlementaire de grande qualité de notre collègue Stéphane Piednoir et du député Jean Luc Fugit, pour le compte de l’Opecst. De nombreuses consultations publiques ont également pu être menées avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Afin d’assurer une pleine maîtrise industrielle, et des standards de qualité et de sûreté au plus haut niveau imaginable dans ce contexte, le Gouvernement a fixé quatre objectifs qui sont autant de principes ayant ayant guidé l’examen de ce texte : l’amélioration de l’efficience des procédures ; l’indépendance de l’autorité par rapport aux exploitants nucléaires et au Gouvernement ; une transparence renforcée vis à vis du public ; l’amélioration de l’attractivité des métiers. Le 31 janvier dernier, nous avons entamé en commission l’examen du projet de loi. La plupart des cinquante sept amendements adoptés concernent les articles 1 à 5 sur l’organisation de la nouvelle autorité. de ces modifications visent à apporter des précisions afin de répondre aux inquiétudes exprimées, notamment concernant la séparation entre les activités d’expertise et de décision au sein de la future autorité, ainsi que sur la publication des avis d’expertise. Notre commission a également introduit au sein de la future autorité une commission d’éthique et de déontologie composée de personnes extérieures qualifiées, comme cela existe actuellement pour l’IRSN. Elle sera chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, d’en suivre l’application et de prévenir les conflits d’intérêts. Suivant encore une recommandation de l’Opecst, un amendement déposé par les deux rapporteurs, dont je salue le travail, vise à pérenniser l’existence de groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences, dont les modalités de nomination resteront précisées dans le règlement intérieur. En séance, cette version du texte a été largement reconduite. Au regard du calendrier, trois points nécessitent une attention particulière dans le contexte d’une activité démultipliée le respect de l’engagement d’un rattrapage des salaires des salariés et contractuels publics ; l’accompagnement des changements majeurs dans les procédures de travail, pour les 500 fonctionnaires et contractuels de droit public de l’ASN et les plus de 1 600 salariés de droit privé de l’IRSN, dans une configuration inédite pour une autorité administrative indépendante ; la mise en œuvre claire des dispositions sociales qui figurent dans le projet de loi. Le groupe RDPI salue la plupart des évolutions intervenues par voie d’amendements et se prononcera majoritairement en faveur du projet de loi et du projet de loi organique. La parole

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, un an après une tentative avortée de fusion brutale et cavalière de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire menée à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, nous sommes réunis aujourd’hui afin de nous prononcer sur la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire dans notre pays. Durant cette année, que s’est il passé ? L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a remis un rapport dont la qualité est indéniable, mais où l’examen d’un scénario d’un renforcement du système dual actuel demeure insuffisant pour un examen complet et une décision claire sur l’avenir de la gouvernance de la sûreté nucléaire. À cela s’ajoute l’absence totale d’audition ministérielle au sein de nos commissions respectives de l’aménagement du territoire et du développement durable, et des affaires économiques. Cela a d’ailleurs été rappelé avec conviction et justesse par la présidente Dominique Estrosi Sassone en ouverture des débats, mercredi dernier. Les lacunes évoquées ont motivé le dépôt puis le vote d’une question préalable et d’une motion de renvoi en commission avec nos collègues du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky et du groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Cette démarche peu commune est le symbole parmi d’autres du parcours législatif chaotique et précipité de ce texte.

C’est un parlementaire qui est né, qui a grandi et qui vit dans un département façonné par l’industrie nucléaire comme aucun autre en France qui vous le dit aujourd’hui. De la production d’électricité au retraitement des déchets, les milliers d’ouvriers de la presqu’île du Cotentin ont toujours cultivé une haute opinion de cette filière d’excellence. C’est bien là le cœur de notre opposition. Loin d’être raisonnée, cette réforme est à rebours de l’histoire du nucléaire français. Elle est marquée du sceau de la précipitation, une précipitation nécessairement mauvaise conseillère lorsqu’il s’agit de la sûreté d’une industrie non conventionnelle, plus encore quand celle ci est à la croisée des chemins d’une relance sans précédent. Cette précipitation, puisque la fusion doit impérativement être effective au 1 janvier 2025, serait justifiée par la quête d’une fluidité présentée comme indispensable à la réussite de la relance de la filière nucléaire. Or à aucun moment du débat parlementaire, y compris lors de l’audition du président de l’ASN, pourtant lui même favorable à la réforme, cette fluidité ne sera apparue comme garantie par la fusion. Elle est et demeure un vœu pieux. C’est même le contraire qui paraît en découler, avec un aveu presque unanime jusque dans les rangs des partisans de la fusion d’une désorganisation annoncée de la sûreté, au moment où notre pays en a le plus besoin. Alors que le système dual actuel a fait toutes ses preuves, est internationalement reconnu et ne demande qu’à être conforté, alors que nous entrons dans une décennie décisive pour la filière nucléaire avec le développement des EPR2 et des SMR, pouvons nous nous offrir le luxe et courir le risque d’une désorganisation profonde et durable de la sûreté nucléaire ? La réponse est assurément non Nous le disons ici solennellement : il ne peut y avoir de relance de la filière nucléaire sans la confiance de nos concitoyens, et cette confiance ne saurait être possible sans la garantie de la transparence. Nous n’ignorons pas la défiance qui peut habiter l’esprit de nos concitoyens et la façon dont le doute sur la véracité des faits peut s’insinuer en eux quand il s’agit de nos institutions, qu’elles soient politiques, scientifiques ou industrielles. Il nous appartient donc de fatiguer ce même doute par une exigence de transparence sans cesse réaffirmée. Or, avec cette réforme, le compte n’y est pas. Le rejet de nos amendements sur la publication des expertises en amont de la prise de décision ou le refus d’une garantie d’indépendance fonctionnelle pour les personnes chargées de l’expertise dans la future ASNR sont autant de mauvais signaux sur le modèle de gouvernance de la sûreté défendu par le Gouvernement.

Mes chers collègues, nous sommes donc appelés à nous prononcer aujourd’hui sur une réforme dont personne ne perçoit les bénéfices, mais dont chacun identifie les méfaits. Cela a été souligné avec force et à maintes reprises par mes collègues Gilbert Luc Devinaz et Franck Montaugé durant la discussion générale et lors de la défense de nos amendements. Soyons à l’écoute des premiers concernés, les salariés de l’IRSN et de l’ASN. Ils ne s’opposent pas à la fusion par conservatisme, par inertie ou par souci de défendre coûte que coûte le. Leur rejet trouve sa source dans leur travail quotidien au service de la recherche, de l’expertise et de la sûreté nucléaire. Ces femmes et ces hommes sont engagés dans une filière exigeante ; et c’est au nom de cette même exigence qu’ils refusent de voir un modèle de gouvernance efficace être démantelé du jour au lendemain. La multitude des avis négatifs formulés à l’égard de ce projet de loi et ses conséquences non maîtrisées doivent nous interroger. La seule voie envisageable pour la gouvernance de la sûreté est celle d’une décision nourrie par l’apport d’un temps de réflexion long et concerté. Ne cédons pas à l’urgence. Donnons à l’IRSN et à l’ASN les moyens budgétaires de l’ambition d’une relance réussie de la filière nucléaire. Confortons leurs missions pour que la triangulation avec l’exploitant, le premier garant de la sûreté, soit maintenue et renforcée. Confions aux deux entités les ressources financières nécessaires pour attirer et conserver en leur sein les compétences rares. Bref, garantissons leur les moyens adéquats et proportionnés pour faire face à la montée en charge programmée. Mes chers collègues, il n’y aurait pas, d’un côté, l’impérieuse nécessité de la fusion et, de l’autre, la faiblesse du. La seule certitude à ce jour est la désorganisation consécutive d’une fusion menée à marche forcée. Fidèle à son exigence d’un nucléaire sûr, fondé sur l’indépendance de l’expertise, la transparence des instances, le respect des salariés et la confiance de nos concitoyens, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera donc résolument contre cette réforme, non seulement inutile, mais aussi néfaste ! Mes chers

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

le nucléaire dans notre pays est à la fois un objet de fierté et d’indépendance. C’est bien récent ! Les conditions de son examen, de son contrôle, de sa sûreté, nécessitent d’avoir un regard qui soit à la fois le plus large et le plus transpartisan possible.

Quand on assume la poursuite de l’exploitation de cinquante six réacteurs nucléaires, quand on relance la construction d’EPR2, quand on relance des programmes de recherche autour des SMR, quand on a comme ambition la consolidation de l’amont et de l’aval du cycle du combustible, il importe de mettre à niveau notre modèle et de le réinterroger. La dualité entraînait des complexités d’interface inévitables, un risque de partage des compétences au moment où nous en avons besoin, des processus et des outils distincts, sources de lourdeur.

une rédaction permettant de couvrir un champ équivalent à celui du travail d’expertise de l’IRSN, soit plus de 300 avis rendus par an. Je salue également les garanties en matière de transparence sur l’activité d’expertise interne qui se poursuivra au sein de la future autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection.

de donner à notre pays les moyens de réussir la relance de la filière nucléaire, tout en maintenant l’excellence de la sûreté et de la sécurité de nos installations. C’est une relance qui est plébiscitée par nos concitoyens et qui nous est rappelée par l’urgence climatique.

le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur, pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour du droit de répartie,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne suis pas d’accord avec le ministre de l’agriculture quand il dit que les problèmes de l’agriculture remontent à plus de trente Si l’on peut s’accorder sur le fait que les agriculteurs ont connu des situations difficiles depuis la nuit des temps, il n’en reste pas moins vrai que cela s’est démultiplié depuis 2015.

La gauche a beau crier que c’est un problème de revenu et de charge de travail, la réalité, même si cela lui déplaît, est que les agriculteurs ne demandent pas à travailler moins ! Au contraire, ils souhaitent retrouver de la liberté pour continuer de travailler plus pays ! Madame la ministre, dans un « en même temps » schizophrène, vous avez fait mine de comprendre leur problème. Vous avez dressé le bon diagnostic. En revanche, vous vous êtes refusée à trouver les solutions pour y remédier. y remédier. C’est une marque de fabrique de la Macronie : on nomme les problèmes et les erreurs commises – concurrence déloyale, suradministration, injonctions contradictoires, normes abusives, etc. –, mais, « en même temps », on s’acharne scrupuleusement à ne pas les résoudre.

Mais chassez le naturel, il revient au galop ! Dès les barrages levés, les mêmes ministres qui ont accompagné le Premier ministre et soutenu ses déclarations et fait leurs ses constats se relaient tour à tour sur les médias pour apaiser la minorité qui les terrorise. Rien ne va changer Rassurez vous : nous ne reviendrons pas en arrière… Au delà d’être schizophrène, cette méthode est mortifère. Comment nommer parfaitement l’erreur d’une surtransposition exclusivement française, en citant les conséquences de l’impasse à laquelle elle conduit, en comprenant les risques majeurs de concurrence déloyale qu’elle provoque pour nos agriculteurs et les risques de perte de souveraineté alimentaire qu’elle fait courir au peuple français et finir, par lâcheté, à ne rien vouloir changer Ne pas vouloir revenir en arrière se paiera dans les années à venir. Vous en serez comptable ! Je vous le dis, les annonces ne calmeront pas la colère, qui reviendra tôt ou tard. Le mal n’est pas guéri, bien au contraire

Ce que cette crise nous dit, c’est que les agriculteurs ne comprennent pas et ne supportent plus cette stigmatisation, ce harcèlement, cette vindicte qui les accablent et qui ne cessent de s’intensifier. Pour répondre à ce malaise, il faut agir vite et fort autour de trois axes prioritaires : arrêter la stigmatisation, mettre un terme à la et revenir sur les erreurs de surtranspositions normatives. Arrêter la stigmatisation, c’est arrêter cette folie française qui consiste à contrôler les faits et gestes des agriculteurs plus que ceux des dealers que ceux des dealers ! C’est arrêter définitivement cette plateforme de délation phytovigilance, qui finit par être la source déguisée de revenus de ces ONG bien pensantes qui dénoncent le moindre écart, la moindre maladresse de l’agriculteur, et instrumentalisent l’OFB en police religieuse de l’environnement. Toute constatation de cette dernière consécutive à une délation relèvera du pénal, donc sera envoyée au procureur. Lui même, pour éviter l’engorgement des tribunaux, demandera à l’agriculteur censément coupable d’accepter un compromis avec les parties civiles, qui ne sont ni plus ni moins que les ONG ONG elles mêmes ou leurs partenaires, et de payer des dommages et intérêts à celles ci, et tout sera réglé. On voit bien que cela sera sans fin…

qu’il n’agit que par bon sens et parce que l’expérience le lui a appris… Très bien ! Enfin, revenir sur les surtranspositions, c’est accepter de corriger ses erreurs en revenant en arrière. en revenant en arrière. Oui ! Si vous ne revenez pas sur l’interdiction de la cinquième famille des néonicotinoïdes, vous ferez disparaître la betterave en France, car ceux là mêmes qui nous expliquaient disposer de méthodes alternatives – l’Inrae, pour ne pas le citer – ont été incapables de les mettre en pratique. ! Et, après les betteraves que l’on a poussées dans le, dès 2026, ce sera le tour de la pomme et de la poire : lorsque le spirotétramate sera interdit en Europe, Europe, elles aussi seront dans l’impasse. Les Polonais, eux, continueront de produire et d’inonder notre marché, car l’acétamipride, interdit chez nous, restera autorisé chez eux, leur permettant de lutter contre le puceron cendré, qui fait des trous noirs à la surface des pommes.

Votre administration ne fait pas mieux : combien de semaines aura t il fallu pour retrouver la simple méthode d’analyse dans vos laboratoires de l’oxyde d’éthylène, interdit en France depuis 1992 ? Vos contrôles aux frontières se cantonneront quasi systématiquement à un contrôle administratif des certificats d’accompagnement de la denrée et d’un contrôle visuel de celle ci. Pensez vous, en toute honnêteté, pouvoir vendre aux Français que les clauses miroirs vont les protéger ? Non ! Et même si, par miracle, vous arriviez à démultiplier les contrôles sur tous les produits importés, le sucre ukrainien, dont les importations sont passées de 20 000 tonnes il y a deux ans à 700 000 tonnes cette année qui est produit avec des betteraves traitées avec les cinq familles de néonicotinoïdes autorisées chez eux et interdites chez nous, passera la barre du contrôle, car il est impossible aujourd’hui de retrouver et de mesurer moindre trace de ces substances dans le produit fini ! Mettons donc fin à cette fumisterie et à cette naïveté coupable qui consiste à détourner le regard, à ne pas vouloir revenir en arrière et à laisser entrer toujours plus de produits étrangers qui ne respectent pas nos normes ! Très bien ! Arrêtons de vouloir courir après un hypothétique changement de modèle

Ayez le courage de le faire, car c’est à ce prix que vous comprendrez, enfin, le mal être des paysans

Après la grippe aviaire, le manque d’eau, le gel et la sécheresse, cette crise de trop a été à l’origine du grand mouvement de protestation de la profession agricole, qui a démarré dans mon département. Ce malaise général qui s’est exprimé dans notre pays couvait depuis un bon moment déjà. Dans le contexte de la crise ukrainienne et de ses conséquences sur le prix de l’énergie, comment faire face ? Depuis de nombreuses années déjà, l’agriculture française doit supporter un permanent et une multiplication de normes, de surtranspositions et de réglementations en tout genre, qui rendent l’exercice de la profession de plus en plus complexe. Face à cette situation, le Gouvernement a dévoilé une panoplie de mesures de compensation financière destinées à aider les éleveurs les plus touchés, comme le gel du gazole non routier (GNR), ainsi que de nombreuses mesures de simplification administrative. Tout cela va, bien sûr, dans le bon sens, mais je suis certain qu’il faut aller plus loin et amorcer un nouveau virage dans la transformation de notre modèle agricole. Le projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles doit être un excellent véhicule pour changer de cap et donner à notre politique agricole les moyens de retrouver sa première place européenne. Arrêtons le démantèlement de la « ferme France » ! Après quelques années d’observation, nous avons pu constater les dégâts causés par certaines mesures dites « vertes », qui partent parfois d’un bon sentiment, mais s’avèrent, à la sortie, mortifères pour nos exploitants. Oui, il faut diminuer nos épandages de pesticides et optimiser la gestion de l’eau, mais il serait souhaitable que l’on parle plus souvent des progrès réalisés dans ces domaines. L’écologie punitive, qui n’a à la bouche que les mots « interdire » ou « supprimer », n’a plus sa place autour des tables de discussions. Cessons d’écouter les Khmers verts et les adeptes de la décroissance ou de la lampe à huile ! La France a besoin d’une agriculture puissante, qui produit et procure un revenu décent à ses acteurs. L’écologie pragmatique nous enseigne que rendements et objectifs environnementaux ne sont pas incompatibles, à condition d’avoir de l’ambition et de faire confiance à la science, qui va nous ouvrir de nouvelles voies de progrès. J’en profite pour saluer la décision du Parlement européen, qui, le 7 février dernier, a enfin décidé l’autorisation encadrée de l’utilisation des nouvelles variétés de plantes, dites NBT,

en créant des distorsions de concurrence au sein même de l’Union européenne, tout en empoisonnant la vie des agriculteurs à grands coups de tracasseries administratives. Quand l’Europe parlera d’une même voix, nous serons plus crédibles sur les marchés internationaux Que dire des programmes Écophyto ou ? L’agriculture « zéro phyto » relève du fantasme d’incompétents notoires ou de rêveurs ! La diminution de nos consommations de phytos ne relève pas de règles arithmétiques. Il faut d’abord trouver des solutions de remplacement et s’adapter. Cette crise structurelle a aussi révélé, s’il en était besoin, les grandes disparités géographiques de notre agriculture, qu’il s’agisse de la taille des exploitations ou du revenu moyen. Dans un tel contexte, il paraît très difficile d’adapter des textes de loi sans observer un principe de différenciation territoriale. On a bien vu que l’augmentation programmée du GNR n’avait pas les mêmes conséquences financières pour tout le monde ! Il semble souhaitable de revenir à un pragmatisme écologique et administratif, afin d’accompagner de manière efficace la transformation de nos exploitations. Il faudra également revoir la copie en matière de formation et d’installation de jeunes agriculteurs. La profession n’échappe pas à la règle qui touche toutes les entreprises sur notre territoire. Les seuils de rentabilité augmentant, il faudra – plus particulièrement dans notre beau Sud Ouest – procéder à des regroupements de propriétés, afin de pouvoir dégager des bénéfices suffisants et faire face à des investissements de plus en plus lourds. Même si ce modèle n’est pas encore ancré dans les mentalités, il devra être porté par les chambres, qui ont été beaucoup trop timides dans ce domaine. Continuons à agir pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée, dans la suite d’Égalim ! D’ici à dix ans, un tiers des agriculteurs sera parti à la retraite. Facilitons la transmission et le regroupement des exploitations afin de donner aux jeunes qui démarrent l’espoir et les moyens de vivre leur passion pleinement. La France sans ses paysans ne serait plus la France. Agissons ! Il y a urgence. Notre souveraineté alimentaire doit redevenir une priorité nationale. La

M. le sénateur Duplomb me permettra de répondre plus globalement à son propos introductif en conclusion du débat. Je partage, monsieur le sénateur, un grand nombre des constats que vous mettez en avant. Oui, vous avez raison, il n’est plus question de faire de l’écologie punitive. Ce n’est d’ailleurs pas notre ligne ! Notre ligne est de ne pas opposer souveraineté alimentaire et transition écologique et de trouver des solutions pour suivre ce chemin,

La ligne que nous tenons est, d’abord, une politique qui soit fondée sur la science, donc qui investit dans la recherche, dans l’innovation et dans le transfert vers les agriculteurs. Le deuxième enjeu a trait à la dimension européenne.

pas de baisser notre niveau d’exigence, mais tout simplement de permettre aux agriculteurs de se concentrer sur ce qu’ils savent bien faire – produire –, sans se perdre dans le maquis

Monsieur le président, mes chers collègues, permettez moi tout d’abord, madame la ministre, de vous féliciter pour vos nouvelles fonctions gouvernementales.

Il y a néanmoins des fondamentaux, que sont la compétitivité, la souveraineté et la nécessité de produire pour des marchés et des consommateurs.

Premièrement, nous devons œuvrer à faciliter la transmission des exploitations agricoles, car il n’y a pas d’avenir sans renouvellement des générations. Un dispositif d’accompagnement des agriculteurs en fin de carrière doit être mis en place pour simplifier l’installation, notamment des incitations fiscales

Depuis vingt ans, l’agriculture s’est attachée à répondre à de nombreuses attentes sociétales et environnementales, sans qu’on lui donne en parallèle les moyens de demeurer compétitive. Un choc de simplification et une pause dans la prolifération normative s’imposent aujourd’hui. Depuis de trop nombreuses années, la multiplication des normes franco françaises a engendré une forme de distorsion dans la concurrence intra européenne, ce qui a fragilisé notre compétitivité. Nous devons nous en tenir

Madame la ministre, votre prochaine loi d’orientation et d’avenir agricoles devra porter l’ambition du redressement de notre agriculture pour que celle ci redevienne une priorité nationale. Nous serons à vos côtés pour y parvenir. La parole est à Mme la ministre

Le pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, qui a été présenté par le ministre de l’agriculture, Marc Fesneau, le 15 décembre 2023, comporte des mesures fortes que nous allons

madame la ministre, mes chers collègues, alors que les mobilisations se poursuivent, et à dix jours de l’ouverture du salon de l’agriculture, nous voici réunis pour débattre de l’avenir de notre modèle agricole. la colère des agriculteurs ne nous a pas surpris, elle a révélé au grand jour à l’ensemble de nos concitoyens l’ampleur de l’impasse dans laquelle le système actuel nous a conduits.

L’avenir de notre modèle agricole dépend de notre capacité à analyser et à agir sur les causes et les impacts de la trop faible rémunération de celles et de ceux qui nous nourrissent. Pour cela, il nous faut regarder en face les dysfonctionnements de notre modèle agricole et de notre système alimentaire,

Les politiques publiques doivent donc contraindre ces acteurs à jouer leur juste part dans la transition, alors qu’ils en sont aujourd’hui largement absents, la plupart des efforts étant demandés aux seuls producteurs.

comment changer de pratiques, voire de système, quand on ne gagne pas sa vie ? En la matière, le revenu agricole est un préalable nécessaire. Le dernier niveau d’inégalité, tout aussi destructeur pour notre système agricole et alimentaire, est celui qui a trait aux revenus de l’ensemble de nos concitoyens. 16 % des Français déclarent ne pas manger à leur faim et la consommation alimentaire des ménages a chuté de 17 % en un an et demi, la décrue étant particulièrement prononcée chez les plus précaires. Ces inégalités, qui explosent depuis quelques années, conduisent une partie toujours plus grande des consommateurs à se tourner vers des produits de faible qualité, pour partie issus de l’importation, et qui ne contribuent ni à la rémunération des producteurs ni à la protection de l’environnement et de la santé. Le remède à ces inégalités structurantes, madame la ministre, ce n’est pas plus de libre échange, plus de compétition internationale, donc de produits issus du moins disant social et environnemental,

La pause dans le plan Écophyto, les attaques envers l’Anses, le mépris de l’agriculture biologique ne répondront en rien à la question du revenu agricole. Pour garantir l’avenir de notre système et la rémunération de nos producteurs, il nous faut plus de régulation des relations commerciales et des marchés, plus de protection face aux importations de produits ne respectant pas nos normes, plus d’équité dans la distribution des aides, plus d’accompagnement des paysans face aux défis environnementaux. Ce n’est aucunement de l’écologie punitive ! Il nous faut construire l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité, voie tracée par les expérimentations, sans cesse plus nombreuses sur les territoires, de sécurité sociale de l’alimentation. Aussi, madame la ministre, quand votre gouvernement cessera t il d’accélérer dans la mise en œuvre de ce système qui appauvrit la grande majorité des agriculteurs aux dépens de notre environnement et de notre santé ? Attendrez vous l’extinction du dernier insecte et du dernier oiseau des champs ? Attendrez vous l’implosion de notre système de santé ? Changer d’indicateur ne change pas la réalité ! Quand cesserez vous de tendre l’oreille à la fabrique du doute ?

nous concilierons souveraineté alimentaire, défense du revenu des agriculteurs et ambitions écologiques et climatiques, non pour le bien de l’Europe ou de la planète, mais pour le bien des agriculteurs et des Français

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nos paysans lancent actuellement un cri de détresse qui est révélateur d’une profonde inquiétude ; celle ci doit nous amener à traiter ce qui constitue le cœur du problème, à savoir le prix payé aux producteurs et le poids des normes qui s’appliquent au monde agricole. Voilà plusieurs années que nous assistons à des mutations profondes de notre modèle agricole – de modèles agricoles. Ces mutations sont aussi le reflet des attentes parfois contradictoires que l’on adresse aux acteurs de la terre agriculteurs gardiens des paysages et animateurs de la ruralité, agriculteurs chefs d’entreprise, agriculteurs 2.0, administrateurs, comptables, ingénieurs, gardiens de la biodiversité et de la sécurité alimentaire : la liste n’est pas exhaustive. Ces mutations sont connues et documentées. politique agricole commune (PAC) et de la banalisation de l’agriculture, qui ont eu un impact sur le revenu agricole, devenu très hétérogène et dépendant des fluctuations des marchés. Dans le même temps, la concentration des autres maillons de la filière agroalimentaire a exercé une pression insoutenable sur le revenu de l’ensemble des agriculteurs, qui bientôt des aides que de leur travail. L’agrandissement des exploitations et l’augmentation de l’intensité capitalistique qui en découle posent la question de la transmission : un agriculteur souhaitant s’installer doit investir bien davantage qu’il y a trente ans pour reprendre une ferme. De même, la prépondérance des formes sociétaires en lieu et place de l’exploitation individuelle et l’apparition d’une agriculture de firme ont généré une augmentation du travail salarié permanent non familial ainsi que l’apparition de nouvelles formes de travail. Le vieillissement de la population agricole risque de compromettre notre sécurité alimentaire, alors même que nous avons perdu 100 000 exploitations en dix ans. Le changement climatique le stress hydrique nous interdisent aujourd’hui d’opposer l’agriculture et la transition écologique. Les agriculteurs, premières victimes du réchauffement climatique,

aux risques environnementaux et sanitaires, à la concurrence déloyale et au dumping social. Comment réussir la transition vers un modèle agroécologique permettant à chacun de se nourrir sainement ? Comment garantir un juste niveau de rémunération, un juste partage de la valeur ? Ces questions se posent alors que, dans le même temps, l’Union européenne s’est engagée dans un processus de négociation de traités de libre échange qui ne répondent ni à nos exigences sanitaires ni à nos exigences sociales, et ce sans ratification par les parlements nationaux. le même temps, 80 % des fonds de la PAC sont alloués aux 20 % des agriculteurs les plus riches, qui pratiquent l’agriculture intensive. Dans le même temps, la stratégie européenne « de la ferme à la table et la PAC n’incluent aucune dimension sociale qui garantisse le respect des droits sociaux et la santé des travailleurs de la terre. Dans le même temps, enfin, les avancées contractuelles permises par les lois Égalim 1 et 2 ont déçu les agriculteurs et eu pour seul mérite d’avoir fait connaître davantage les coûts de production, sans faire respecter pour autant Nous le redisons avec force : seule une remise en cause profonde des rapports de force dans la chaîne de valeur peut véritablement changer la donne. Il faut, à cet effet, que l’État et les agriculteurs eux mêmes interviennent directement dans la formation des prix et des marges

dans le même temps, de restaurer une administration déconcentrée dotée de moyens au service des agriculteurs. Nos propositions sont un préalable indispensable pour freiner les stratégies de délocalisation agricole

Pourquoi a t il fallu que les tracteurs sortent des champs pour que l’on comprenne enfin la détresse des paysans ? Pourquoi, dans ce pays, faut il toujours attendre que la fronde gronde ? Nous ne découvrons pas les bas revenus, la disparition des exploitations, la baisse des transmissions, la lourdeur administrative, les crises climatiques, sanitaires, économiques

nous de ces visières qui nous empêchent d’avancer et abandonnons ces réponses qui nous font tourner en rond ! Réjouissons nous de cette agriculture plurielle et attaquons nous à la vraie question : quel avenir pour notre agriculture ? Partons d’un constat positif : nous avons l’agriculture la plus saine du monde et nos agriculteurs se sont engagés dans des modèles vertueux, car ils sont responsables – et les Français l’ont bien compris. Pourtant, ils ne bénéficient pas de revenus qui soient à la hauteur des services rendus à notre nation et à notre souveraineté.

? Le signal est désastreux tant pour la protection de l’environnement que pour celle de la santé publique ; il va à rebours de nos politiques agricoles et de la transition écologique à laquelle notre agriculture ne pourra se soustraire.

Allez vous enfin comprendre que, pour réussir notre transition, il faut encourager les agriculteurs à s’engager dans la démarche des paiements pour services environnementaux de possibilités qui, une fois mises en place, seraient valorisées par une rémunération au minimum équivalente au coût lié à la perte de productivité induite par ces mesures. Telle est la seule façon de répondre à la particularité de chaque territoire et au besoin d’une agroécologie cohérente, tout en permettant à nos agriculteurs Coupe feux, haies, irrigation raisonnée, restructuration du sol, cépages résistants… : si nos modèles de production doivent évoluer, cela ne pourra se faire de manière uniforme, nos territoires étant marqués par des différences structurelles et climatiques notables.

Faisons le pari du consensus et de la vision de long terme afin de redonner de l’attractivité aux métiers de l’agriculture, d’accompagner et de revaloriser les actifs du monde agricole et agroalimentaire français, d’assurer notre souveraineté alimentaire et de mener la transition agroécologique.

aux exploitants agricoles qui s’engagent volontairement à mettre en place sur leur exploitation des pratiques agronomiques favorables au climat. Ce paiement est découplé, uniforme et versé annuellement sur tous les hectares admissibles de l’exploitation. Tel est par exemple le cas du bonus «

Buis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si tout n’est pas à jeter dans le modèle actuel, il faut bien reconnaître que les manifestations du monde agricole nous obligent. Elles nous obligent à réajuster ce modèle, sur notre sol comme à l’échelle européenne. Si nous voulons demain une France fière de ses paysans et souveraine d’un point de vue alimentaire, nous devons affronter plusieurs défis, du juste revenu à la transmission des exploitations, en passant évidemment par la question des transitions face au dérèglement climatique. Commençons par la question essentielle des revenus. Le constat est sans appel : une partie importante des agriculteurs travaillent pour nous nourrir sans pouvoir eux mêmes vivre lois Égalim, la majorité présidentielle a apporté des réponses. Nous constatons aujourd’hui que le problème vient non pas de la loi, mais de son application, voire de son détournement. Alors, que faire ?

Pour ce qui est de l’Union européenne, il ne faut pas se tromper de combat. À quelques mois des élections européennes, ne cédons pas aux sirènes populistes et europhobes ! La politique agricole commune et ses 9 milliards d’euros sont des acquis que nous devons préserver. C’est à l’échelle européenne que nous parviendrons à développer une agriculture résiliente et souveraine ; c’est en harmonisant les règles que nous encouragerons la coopération européenne et empêcherons les concurrences déloyales. l’échelle européenne est décisive, nous devons d’ores et déjà agir en France pour assurer à nos agriculteurs un meilleur revenu. L’État et les collectivités doivent être exemplaires, par exemple en privilégiant l’achat de produits français en circuit court dans le cadre de la restauration collective.

madame la ministre –, en 1988, on dénombrait 1 million d’exploitations agricoles en France. En 2022, ce nombre a chuté à 380 000. Ce phénomène touche particulièrement l’élevage. En dix ans, la Drôme a ainsi perdu 18 % de ses exploitations, notamment dans les secteurs bovin, porcin et caprin.

sans doute pas un métier qui suppose de travailler soixante dix heures par semaine dans des conditions physiques éprouvantes, pour des revenus modestes, en subissant une inflation d’injonctions administratives et environnementales ! En réalité, la question de l’attractivité est liée à toutes les autres

premier exemple concerne le versement d’aides financières pour les embauches de bergers et d’aides bergers. La période d’embauche s’étend de juin à septembre. L’agriculteur fait l’avance et la subvention compensatrice est versée non pas dans les semaines suivantes, mais douze mois plus tard. Pourquoi un tel décalage ? Les professionnels ont du mal à le comprendre et une telle situation n’incite pas à poursuivre cette activité. Le second exemple, toujours relatif aux éleveurs, concerne l’indemnisation des pertes de brebis en cas de prédation. prédation. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une attaque de loup n’est pas toujours synonyme de carnage. Il est souvent des attaques qui, plus discrètes et plus pernicieuses, ne causent qu’une ou deux pertes par nuit. En fonction de la taille du troupeau, il n’est pas toujours facile de les recenser. Le groupement pastoral

Alors que l’élevage décline, comment repenser le système d’accompagnement des éleveurs ovins pour qu’aucune perte ne se retrouve dans un angle mort de l’indemnisation ? Je pense également aux louvetiers, dont les conditions de travail et l’indemnisation des déplacements pourraient être améliorées. Tous ces exemples montrent, parmi tant d’autres, que les normes ne facilitent pas toujours le quotidien de nos agriculteurs. Enfin, il reste à relever un défi majeur, pour lequel les agriculteurs seront des alliés irremplaçables : celui des transitions face au dérèglement climatique. Comme l’écrivent Erik Orsenna et Julien Denormandie dans leur récent ouvrage, la question de fond est la suivante : comment nourrir sans dévaster ? Comment nourrir 68 millions de Français sans détruire les sols, la biodiversité, notre santé, mais également notre patrimoine, notre savoir faire et ce qui fait de la France le pays de la gastronomie ? Des irrigateurs de Mésopotamie aux éleveurs porcins d’Ausson, dans le secteur de Die, les agriculteurs sont l’une des professions les plus anciennes de notre civilisation. Ils ont démontré leur capacité à s’adapter ; mais nous devons les accompagner plutôt que les accuser et les délaisser. N’opposons pas les modèles d’agriculture et favorisons la coopération ! C’est ainsi que nous pourrons créer un modèle agricole souverain et plus juste. Madame la ministre, à la veille de la Saint Valentin, la politique devrait peut être s’inspirer de la symbolique de cette fête : dire que l’on aime nos agriculteurs, c’est bien, mais le leur prouver, c’est mieux

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, souveraineté et autonomie alimentaire des territoires, renouvellement des générations, agriculture rémunératrice et adaptée au dérèglement climatique, transition agroécologique au sein du groupe socialiste du Sénat, nous sommes parfaitement conscients des nombreux enjeux auxquels doit faire face notre modèle agricole. Nous débattons aujourd’hui de l’avenir de ce modèle, et nous aurons certainement à examiner dans quelques semaines une loi d’orientation agricole, car – oui ! – il est indispensable de fixer un cap clair et précis pour les années à venir. L’avenir, madame la ministre, passera par une formation agricole à la hauteur des nouveaux enjeux. Au delà de la création d’un bachelor agricole, qui viendra directement concurrencer des licences professionnelles existantes, il est indispensable d’améliorer et de valoriser les qualifications des enseignants par la création d’une agrégation propre,

de l’enseignement conduit naturellement à celui de l’installation, dans un contexte de renouvellement des générations. L’idée d’un guichet unique par département peut être positive, mais elle nécessitera une grande coordination avec les autres instances – tout particulièrement les chambres d’agriculture –, et surtout un cadre ouvert donnant la priorité à l’installation, y compris des personnes non issues du monde agricole.

Les agriculteurs veulent avant tout vivre de leur production sans dépendre d’un système de compensation permanente et de réaction aux différentes crises. En dépit des lois Égalim, l’éternelle question de la répartition de la valeur entre les industriels, la grande distribution et les agriculteurs demeure bien, hélas

et des sanctions. Pour ce qui concerne les aides PAC, nous considérons que le logiciel est également à revoir, et ce d’autant plus si l’élargissement de l’Union européenne se confirme. La France doit avoir le courage politique de défendre un plafonnement des aides PAC pour induire davantage de justice sociale dans ce système, comme l’a fait l’Espagne. Surtout, elle doit proposer une véritable modulation des aides entre les filières en fonction de l’évolution des cours, comme c’est le cas aux États Unis avec les aides contracycliques. Ce sujet me conduit à évoquer la nécessité d’accompagner les agriculteurs pour assurer la transition de notre modèle. Ayant été agriculteur pendant plus de vingt ans, j’ai bien conscience que les injonctions ne sont pas toujours faciles à accepter. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics doivent se positionner comme des accompagnateurs de la transition agroécologique. est indispensable pour la santé des agriculteurs, pour leur activité, qui est très fortement affectée par le dérèglement climatique, et pour la préservation de la biodiversité. Le succès des mesures agroenvironnementales et le nombre d’installations en bio attestent cette volonté de changement, mais il faut que l’État

La question du bien être des paysans est également centrale. Bien que le dispositif du crédit d’impôt en faveur du remplacement temporaire ait été amélioré ces dernières années, nous appelons de nos vœux une prise en charge à 100 %, qui paraît pleinement justifiée au regard du rôle nourricier joué par les agriculteurs. Enfin,

et de la fermeté de la part de la France, afin que ne soit pas accepté un accord dangereux pour nos agriculteurs et pour les consommateurs français et européens. Mes chers collègues, l’avenir de notre modèle agricole passera par une prise par des exploitations à taille plus humaine, plus facilement transmissibles, permettant une juste rémunération et favorisant le bien être des agriculteurs, par une révision de la PAC dans le sens de davantage d’équité, et surtout par un accompagnement des agriculteurs vers une indispensable transition. Madame la ministre, j’espère que vous entendrez avec sérieux nos différentes propositions. La parole

sont l’un des enjeux de l’attractivité des métiers et de la politique que nous voulons mener pour favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre nation a une longue histoire d’agriculture prospère. Qui a oublié la phrase : « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France » ? Elle date un peu et, malheureusement, les temps ont bien changé. La France n’est plus ni le grenier à blé de l’Europe ni le deuxième exportateur mondial… Il y a cinquante ans, nous comptions plus de 1,2 million d’exploitations agricoles ; il y en a aujourd’hui un peu moins de 440 000. Sénateur depuis trois ans, j’ai déjà assisté à de nombreux débats relatifs à l’agriculture, voté un certain nombre de textes, entendu de grandes annonces dont la concrétisation allait changer le monde agricole ; et pourtant, ce secteur demeure durablement en crise. Je vous le rappelle, mes chers collègues, 20 % des agriculteurs français vivent sous le seuil de pauvreté. Leurs revendications ne semblent pas irréalistes : ils souhaitent juste pouvoir vivre correctement de leur travail

Finalement, le Gouvernement a attendu que la marmite déborde pour proposer un avant projet quasi vide et prendre des décisions sous la pression. L’annulation de la hausse du GNR est elle vraiment la réponse aux attentes du secteur ? Ce n’est pas certain du tout, et vous le savez, aux problèmes de l’agriculture est multiple. L’avenir de notre modèle agricole est lié à des défis tels que le renouvellement des générations, la fiscalité des transmissions, les charges et la fiscalité qui pèsent sur les agriculteurs, la compétitivité internationale, la transition écologique. Le vieillissement de la population agricole en France est un défi majeur. Et la transmission des exploitations se heurte souvent à des problèmes fiscaux qui peuvent décourager les jeunes agriculteurs. Les droits de succession sont un frein important à la transmission des exploitations agricoles : les héritiers, souvent des membres de la famille, ont parfois du mal à assumer les coûts fiscaux élevés associés à la transmission. peut conduire à des ventes ou à des situations financières difficiles. La question de la fiscalité des transmissions est donc cruciale pour assurer le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations. Les agriculteurs font aussi face à des charges importantes liées aux coûts de production, à l’achat de matériel ou aux coûts salariaux. De surcroît, la fiscalité agricole, qui est complexe, les soumet à une multitude de taxes et autres prélèvements. La dernière source de compétitivité de nos agriculteurs est malheureusement la baisse de leurs revenus, à défaut de celle de leurs coûts de production… Les revenus ne doivent pas être la variable d’ajustement de la compétitivité

de la République plaidait pour « la montée en qualité, la montée du bio » : les produits français moins compétitifs devaient monter en gamme pour atteindre des marchés de niche qui seraient plus rémunérateurs. « en même temps », il allait ouvrir le marché aux produits étrangers de milieu de gamme, mais beaucoup moins chers. Cette politique agricole à deux faces se révélerait une impasse

Les agriculteurs français doivent être en mesure de produire de manière compétitive sur le marché mondial, tout en respectant les normes environnementales et de qualité. Oui, il est possible de protéger notre agriculture des distorsions de concurrence qui ont cours au sein de l’Union européenne et avec le reste du monde Un texte a été adopté au Sénat, l’année dernière, en ce sens ; depuis, il semble s’être perdu dans la tuyauterie de l’Assemblée nationale… Enfin, la transition écologique vers des pratiques agricoles plus durables et respectueuses de l’environnement est un véritable enjeu. Les incitations fiscales visant à encourager les agriculteurs à adopter de telles pratiques peuvent jouer un rôle crucial dans cette transition. Préférons l’usage de la carotte à celui du bâton L’avenir du modèle agricole français dépend de notre capacité à relever ces défis avec détermination, en délaissant les postures politiciennes. Vous avez eu de nombreuses possibilités, ces dernières années, d’améliorer le quotidien de nos agriculteurs ; pourtant, madame la ministre, vous n’avez jamais utilisé les véhicules législatifs

dans des surtranspositions mortifères qui, si elles peuvent apparaître louables sur le plan écologique, conduiront à une baisse de notre production et à une augmentation de nos importations en provenance de pays qui ne sont pas aussi vertueux que le

Au chapitre des contraintes, toujours, il convient d’aborder le sujet du plan Eau. Là aussi, madame la ministre, il faut agir et sortir des carcans administratifs ! Le réchauffement climatique nous met devant le fait accompli : certaines zones de notre pays ne pourront plus être cultivées comme elles le sont aujourd’hui. Il faut apprendre à vivre avec cette réalité, sans déni,

En zone industrielle ou artisanale, par exemple, la présence d’un parking ou d’un espace trop peu fréquenté engendre à elle seule l’application d’une distance de non traitement, alors même que le risque sanitaire est inexistant. Ne serait il pas opportun de mettre en place une nouvelle classification pour répondre à ce problème concret et rendre ainsi des terres à l’agriculture ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le monde agricole français et européen traverse une crise profonde. Le mécontentement des agriculteurs est immense. Pour leur part, les viticulteurs

Espérons que les démarches entreprises auprès de la Commission européenne permettront de sortir très vite du carcan des règles et de la moyenne olympique. Nous attendons encore des réponses concernant l’aide au stockage privé, le déploiement de l’année blanche bancaire et le rééchelonnement des prêts garantis par l’État (PGE) pour les caves coopératives. Nous réclamons des actes très forts et courageux pour nos viticulteurs en détresse. Autre source de mécontentement : la lavandiculture. Comment comprendre que le reliquat de 4 millions d’euros, sur les 10 millions d’aides votées par le Sénat, n’ait toujours pas été versé aux lavandiculteurs ? Quant à la filière française de cerises de bouche et d’industrie, elle est en péril absolu

le mot d’ordre du mouvement de protestation du monde agricole que notre pays vient de connaître est à mon avis loin d’être un slogan anecdotique. Une partie non négligeable des revendications des agriculteurs a tourné autour de l’idée de simplification administrative, une nouveauté marquante de ce mouvement. Autant vous le dire d’emblée : en tant que président de la délégation sénatoriale aux entreprises, cela ne m’a pas réellement surpris ! Le secteur agricole est le plus touché par cette frénésie normative, ce réflexe de tout régler par la loi, le décret et l’arrêté, ce même réflexe qui obère notre potentiel productif. Quel secteur, madame la ministre, connaît des contrôles aussi fréquents que la profession agricole ? des critères d’éligibilité aux dispositifs surfaciques de la PAC, tels que la vérification du couvert déclaré sur les parcelles, fait l’objet d’observations par relevé satellitaire tous les trois jours : tous les trois jours, vous ne rêvez pas

C’est l’histoire du fameux ratio de prairies permanentes ou des règles applicables aux haies, qui pénalisent les bons élèves pour s’être engagés dans des pratiques vertueuses. À force de sanctuariser ces dernières, les agriculteurs vont ils bientôt devoir se cacher quand ils les mettent en œuvre ?

Parce que les normes sont en apparence non coûteuses, elles sont souvent préférées aux subventions ou aux taxations. Pourtant, leurs effets distorsifs sur l’économie sont nombreux et souvent pires que ceux de la fiscalité parce que les normes favorisent la recherche de rente, parce qu’à force de tout faire reposer sur la norme et sur la contrainte, on décourage les motivations intrinsèques et la volonté de bien faire. Soyons clairs : la simplification administrative et le toilettage normatif ne signifient pas l’abandon de toute ambition en matière environnementale ni l’imposition d’un modèle agricole unique mais il est temps de faire un peu de ménage dans nos codes. À cet égard, reconnaissons le, les annonces du Premier ministre vont plutôt dans le bon sens, notamment sur le curage des cours d’eau, les délais de recours contre les projets agricoles ou les projets de gestion de l’eau de l’eau et les seuils d’évaluation environnementale dans l’élevage. Mais force est d’admettre que certaines zones d’ombre subsistent. Par exemple, on ne comprend pas très bien en quoi pourra consister concrètement l’unification du régime applicable aux haies.

Quant à nous, parlementaires, nous devrons nous montrer vigilants lors de l’examen des textes à venir sur la simplification et sur le renouvellement des générations, car il n’est pas rare que des intentions de simplification se traduisent par des réalisations en définitive encore plus complexes Or je suis persuadé que l’avenir de notre modèle agricole dépend avant tout de notre capacité à libérer les initiatives individuelles et à faire confiance à nos 400 000 agriculteurs, notamment aux plus jeunes d’entre eux, pour qu’ils inventent leur propre avenir. La parole

au traitement des contentieux relatifs aux projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installation d’élevage, ou encore à la sécurisation juridique des travaux agricoles et forestiers. Il arrive parfois que

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les agriculteurs ne sont plus sur les routes, ils sont retournés travailler, mais nous savons tous ici que rien n’est réglé. Les paysans français restent enserrés dans le double corset de réglementations nationales contraignantes et de stratégies européennes décroissantes. l’échelon national, l’empilement des lois, des normes et des décrets contraint notre pays, pourtant premier pays agricole d’Europe, à importer la moitié de ses fruits et légumes. À titre d’exemple, dans mon département, en Loire Atlantique,

la Commission européenne est alors intervenue pour demander sa suspension, dans l’attente de la mise en œuvre d’une loi à l’échelon européen. Et l’administration française a donc publié un troisième décret, en juin dernier ! Trois décrets,

En moins de cinq ans, quatre études ont été menées pour évaluer les conséquences de cette stratégie agricole : une étude du département américain de l’agriculture,

Toutes ces études résonnent comme autant de signaux d’alerte que vous avez ignorés. Elles convergent pour souligner trois risques majeurs de la stratégie à l’horizon 2050. Le premier risque, c’est une baisse globale de la production agricole européenne, de l’ordre de 12 % à 15 % selon les études. Le deuxième, c’est une forte hausse des prix des produits agricoles, évaluée entre 12 % et 17 %.

Nous allons tout droit vers « une alimentation à deux vitesses, avec du local pour les riches, et des produits importés pour les pauvres », selon les termes du think tank bruxellois. Enfin,

que les États membres puissent à la fois poursuivre ce processus d’accompagnement des filières agricoles dans leur transition, mais également lutter contre la concurrence déloyale d’autres pays. Tel est l’enjeu des clauses miroirs et des différentes négociations que nous menons avec

Si vous faisiez campagne autre qu’électorale, vous auriez senti venir le mouvement de contestation, le ras le bol actuel. Ce mouvement n’est pas le fruit d’un sentiment ni ne procède de la défense de privilèges, il est le dernier cri du cœur de la paysannerie française, qui ne veut pas mourir. Il n’y a plus de trésorerie dans les caisses des fermes. La propriété réelle se réduit comme peau de chagrin : les matériels appartiennent à la banque, tandis que l’État applique une imposition abusive sur les transmissions d’exploitation. En France, l’agriculture est nourrie par la générosité de ses nappes phréatiques, mais elle est asséchée par une chape de plomb administrative et pseudo environnementale. Notre pays a tout ce qu’il faut pour produire, mais vous faites le choix, madame la ministre, par la voix de vos députés européens et aux côtés de la Commission européenne, de la déproduction En trente ans, l’écolo gauchisme, systématiquement suspicieux à l’égard de nos entrepreneurs, a eu raison de notre civilisation paysanne. À Bruxelles comme à Paris, nos gouvernants ont ligoté les paysans à grand renfort de normes, de restrictions, de contrôles satellitaires et, désormais, de quotas de jachères et de hausse de la taxe sur le GNR, tout cela pour donner libre cours aux traités de libre échange avec l’extérieur de l’Union européenne, à la concurrence déloyale à l’intérieur par la surtransposition et à la dépossession des petits fermiers par les agro industriels. L’agriculture a connu le plus grand plan social de ces trente dernières années. Nous sommes passés de 1,6 million d’agriculteurs dans les années 1980 à moins de 400 000 aujourd’hui. Parmi ces dépossédés, combien ont perdu la vie au champ, au champ d’honneur de la détresse et de l’épuisement ? Pour faire face à l’urgence, il faut impérativement reporter les échéances bancaires des agriculteurs sur l’année en cours et refuser la hausse de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour prélèvement sur Appliquons la politique de la chaise vide à Bruxelles pour récupérer les 11 milliards d’euros que nous versons à la Commission sans en revoir la couleur. Il y a des milliards pour l’Ukraine ;… Parlez en à Jordan Bardella… … il en faut d’abord pour la survie de nos paysans Madame la ministre, depuis mai 2022, l’intitulé du ministère de l’agriculture s’est vu adjoindre l’objectif de « souveraineté alimentaire ». En même temps, le nouveau chef du Gouvernement prône la souveraineté européenne à Berlin. Doxa et paradoxe : aucune cohérence, aucune émancipation à l’égard de la ! Vous jouez la montre électorale, mais les paysans sont de retour, car ils ont compris que vous les aviez trompés. Et pourtant, s’il existait une vision pour l’avenir de notre modèle agricole, elle anticiperait

Parlons d’avenir, madame la ministre : que pensez vous, sur les plans sanitaire et environnemental, des viandes de synthèse, dont le ministre de l’économie a fait la publicité ? Madame la ministre, vous qui faites partie d’un gouvernement en marche permanente et qui n’êtes donc attachée à aucun territoire, vous qui, où que vous soyez, en Corrèze ou au Zambèze, ne considérez la terre des hommes que comme une simple parcelle du marché mondialisé, soyez convaincue qu’une large majorité de Français enracinés restent très attachés au triptyque « pays, paysans, paysages », indissociable de la devise « liberté, égalité, fraternité »… à laquelle

Monsieur le président,

Dans les semaines et mois à venir, je serai mobilisée pour valoriser notamment cette dernière dimension. Je voudrais plus particulièrement m’arrêter quelques instants sur quatre chantiers sur lesquels nous souhaitons, Marc Fesneau et moi même, orienter prioritairement notre action.

Il s’agit de former plus, mais aussi de former différemment, à des métiers qui évoluent sans cesse et qui sont marqués par une forme d’hybridation des compétences requises.

Vous aurez à vous saisir de certaines de ces mesures lors de l’examen du projet de loi : je pense à la rénovation des missions de l’enseignement agricole, à l’institution d’un bachelor agro ou à la création de contrats locaux qui permettront de relancer ou d’ouvrir des classes formant aux métiers de l’agriculture dans nos territoires. Le deuxième défi, c’est celui des transitions agroécologique et climatique. Le Sénat a voté en décembre dernier des moyens inédits pour notre agriculture ; en particulier, cette année, 1,3 milliard d’euros supplémentaires sont dédiés à la planification écologique. Je le dis sans détour

poursuivre nos efforts en matière de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, en gardant en tête ce principe essentiel, « pas d’interdiction sans solution », ce qui suppose évidemment des investissements importants dans la recherche et développement.

Le Premier ministre a pris une décision forte en annulant la hausse de la fiscalité prévue sur le GNR : celle de maintenir les dispositifs de compensation qui y étaient liés. Ceux ci font écho à des propositions formulées ici même, comme le régime du microbénéfice agricole ou la déduction pour épargne de précaution. nous allons plus loin, en enrichissant le projet de loi qui vous sera présenté d’un volet de simplification visant, par exemple, les projets de stockage d’eau ou d’élevage. En effet, libérer les agriculteurs de normes devenues superflues ou contradictoires, c’est leur donner plus de compétitivité, comme vous avez été nombreux à le souligner. Enfin, pour garantir la cohérence de notre action dans ces trois directions – renouvellement des générations, transitions, compétitivité – et permettre à nos producteurs de mener ces grandes transformations, nous avons besoin d’un cadre international et européen qui protège de la concurrence déloyale. Le Premier Le Premier ministre a réaffirmé la volonté de la France d’œuvrer en ce sens. À court terme, une clause de sauvegarde sera mise en place sur les produits agricoles contenant des résidus de thiaclopride et, sur le plus long terme, nous soutiendrons la création d’une force de contrôle sur la concurrence déloyale en agriculture aux frontières de l’Union européenne.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat demandé par notre groupe Les Républicains, lancé par notre collègue Laurent Duplomb, est un débat essentiel pour toute société qui, comme la

le 1 octobre 2017, sur le parvis de la gare Saint Charles, Mauranne, 20 ans, étudiante en médecine, et Laura, 21 ans, élève infirmière, se voyaient ôter la vie

n’ont fait que me conforter dans mes convictions : les transports n’échappent ni au terrorisme ni aux actes de délinquance. Bien au contraire, les transports en commun démultiplient Nous le savons, le risque zéro n’existe pas ; à cet égard, je n’intenterai aucun procès en inaction – et surtout pas à vous, monsieur le ministre, qui venez de prendre la tête de ce beau ministère.

J’appelle à une sérieuse prise de conscience de la part de tous – et je tourne mon regard vers les collègues qui siègent du côté gauche de notre hémicycle. La réalité est implacable et ne saurait souffrir, mes chers collègues, que l’on se raccroche encore, malgré des faits de plus en plus nombreux et de plus en plus violents, à des espérances angéliques et à des clichés dépassés. Je vous propose plutôt que nous nous posions la question suivante : comment pouvons nous, en tant que législateurs, inciter les usagers à privilégier de manière massive le recours aux transports en commun, si certains d’entre eux – je pense en particulier aux femmes – évitent ces réseaux en raison de l’insécurité, comme c’est le cas aujourd’hui ? Très bien ! Bravo ! Ne vous laissez pas aveugler par une certaine idéologie d’un autre temps Je vous propose simplement d’améliorer utilement l’arsenal de sécurité dans les transports, qui est aujourd’hui à bout de souffle. C’est une urgence au regard du contexte, car la police nationale, dont je salue le dévouement, ne peut être partout. Et les transports sont par nature vulnérables à la menace terroriste, aux violences sexuelles, aux atteintes aux personnes et aux biens, à la fraude… Pour que chacun prenne bien la mesure de la réalité, voici quelques chiffres : en 2022,

Il est de notre devoir d’améliorer la sûreté dans les transports collectifs par des actions de prévention et de répression. C’est là tout l’objet de la proposition de loi que nous discutons aujourd’hui ; je tiens d’ailleurs à remercier Bruno Retailleau, qui a souhaité l’inscrire à l’ordre du jour.

des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Les constats ont été limpides, partagés. Sans que cela remette en cause les prérogatives des forces de sécurité intérieure, les agents de la

Leur but n’est en aucun cas d’attenter aux libertés, mais, au contraire, de les préserver, en protégeant les usagers, les conducteurs et les agents – qui sont tous, je le rappelle,

présent sur place un officier de police judiciaire, l’individu appréhendé doit être laissé libre avec ses objets. Ces mêmes agents ne peuvent interdire à une personne d’entrer en gare alors même qu’elle a un comportement dangereux à l’extérieur.

selon cinq principaux axes. Elle vise, premièrement, à étendre les prérogatives des services internes de sécurité des opérateurs de transport que sont la Suge et le GPSR, en renforçant leur faculté à procéder à des palpations préventives et en créant une véritable interdiction d’entrée en gare. deuxièmement, d’améliorer le continuum de sécurité dans les transports en pérennisant l’utilisation des caméras piétons sur la voie publique ou en permettant à la police municipale de mieux accéder aux réseaux Le troisième axe consiste à recourir davantage à la technologie, notamment au traitement algorithmique, pour répondre aux réquisitions judiciaires. Le quatrième est de lutter efficacement contre la fraude par un meilleur recouvrement. Sur 2,4 millions de procès verbaux dressés par la SNCF, représentant un montant de 275 millions d’euros, seuls 22 millions d’euros ont été recouvrés dans les délais légaux. Voilà qui n’est plus acceptable Cinquièmement, enfin, nous devons mieux réprimer les délits. Je propose une extension du délit d’habitude afin de punir sévèrement aussi bien les récidivistes de la fraude que ceux qui récidivent dans la commission d’incivilités telles que cracher, uriner, souiller, détériorer, ! Soyons clairs sur ce que nous voulons mettre en place : tu menaces la quiétude ou la sécurité des voyageurs, tu seras désormais sanctionné ! Je propose également une interdiction de paraître, pour qu’enfin les multirécidivistes du harcèlement sexuel soient empêchés de pénétrer dans les réseaux de transport. Mes chers collègues, tant que nombre de nos concitoyens éviteront les transports en commun pour des raisons d’insécurité, tous les financements

Je forme ainsi le vœu que nous parvenions collectivement à dépasser nos clivages sur ce sujet. Ce sera – derechef je l’espère – tout le sens de l’arbitrage pris par le Gouvernement et entériné par la conférence des présidents consistant à retenir la procédure accélérée pour l’examen de cette proposition de loi.

insiste, de nourrir la chimère du risque zéro par d’inutiles surenchères sécuritaires – ce serait illusoire. Il faut agir pour une sécurité concrète. en France, à bien des égards, l’histoire du transport en commun et des chemins de fer accompagne celle de la Nation. Traditionnellement, les professionnels du transport s’emparent de la sécurité, et les forces régaliennes de la sûreté. Mais cette séparation des tâches n’a pas résisté à l’épreuve du temps. La gravité de la situation impose un nouveau choc. Notre responsabilité est d’y répondre, non seulement pour endiguer ou réprimer le passage à l’acte délictueux, mais également pour protéger les citoyens usagers ; tel est notre devoir.

Ce texte vise à combler plusieurs lacunes de la législation pénale en vigueur et à octroyer aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF les moyens administratifs, judiciaires et opérationnels indispensables à la sécurisation efficace des transports en commun. Sur le fond, la commission des lois ne pouvait qu’accueillir favorablement cette proposition de loi, qui reprend des dispositions déjà votées par le Sénat, notamment dans les lois dites Savary Leroux globale. Comme j’ai pu le constater au fil des auditions que j’ai menées, elle est le fruit d’une réflexion approfondie, nourrie des observations et propositions des acteurs de terrain que sont la Suge et le GPSR, qui sont en première ligne pour sécuriser nos gares et nos transports en commun. Le législateur a régulièrement renforcé les moyens des acteurs du continuum de sécurité dans les transports, mais il s’est concentré sur la répression de la fraude tarifaire et la lutte contre le terrorisme, sans parvenir à une réponse globale en ce qui concerne la lutte contre les incivilités et la délinquance spécifique aux transports collectifs. Les gares ferroviaires, les stations de métro et de bus, les réseaux ferrés ainsi que les véhicules de transport sont, par nature, vulnérables à différentes menaces : menace terroriste, violences sexuelles et sexistes, atteintes aux biens et aux personnes. Les gares, lieux de passages ouverts, dotés de multiples accès et concentrant une forte densité de population, comme les matériels roulants, espaces confinés et facilement accessibles, sont exposés à des risques de sûreté majeurs.

ciblées pour ces lieux. Cependant, force est de constater que la situation actuelle reste peu satisfaisante, et même paradoxale à certains égards.

Comment expliquer que les agents de la Suge ou du GPSR doivent interrompre la poursuite d’un individu qui, pris sur le fait, s’échapperait en courant en dehors de la gare, où ils ne peuvent intervenir ? Comment expliquer que des défis consistant à monter sur le toit de rames de métro ou de bus en marche ne soient pas délictualisés ? Enfin, je voudrais dire un mot du contexte particulier dans lequel nous légiférons : ces mesures sont rendues d’autant plus indispensables que notre pays s’apprête à accueillir, pendant près de deux mois, les jeux Olympiques et Paralympiques. Cette proposition de loi ne tend pas à bouleverser les équilibres sur lesquels repose notre continuum de sécurité, ni remettre en cause le rôle de chacun. Son objectif principal est d’apporter des réponses

à l’équilibre entre opérationnalité des mesures, garantie des droits et libertés constitutionnels et cohérence du continuum de sécurité dans lequel ces services internes de sûreté s’inscrivent. Nous avons retenu un grand nombre de dispositions : interdiction d’entrée en gare ; peine d’interdiction de paraître dans les transports

d’autres instruments ou techniques moins attentatoires aux droits et libertés existent, nous avons préféré supprimer quatre mesures : la faculté de procéder à des palpations de sécurité de manière inopinée la possibilité de collecter des données sensibles en dehors des cas de flagrance ; le déploiement d’instruments de captation du son au sein des véhicules ferroviaires ; l’intervention sans condition des équipes cynotechniques de la SNCF.

aux amendements de Louis Vogel et Marie Claire Carrère Gée, qui visent à prolonger d’un an l’expérimentation du recours aux traitements algorithmiques pour répondre aux réquisitions judiciaires,

Ces initiatives permettant d’enrichir utilement le texte, j’y serai favorable. Pour ma part, outre des amendements rédactionnels, je déposerai, comme je m’y étais engagée,

ayons trouvé une voie juridiquement robuste sur ce sujet particulièrement important sans pour autant remettre en cause le transport d’objets licites dans les lieux publics que sont les gares. À ce sujet, j’aimerais partager avec vous une réflexion plus générale que je tire des travaux que j’ai menés sur ce texte. Nous touchons ici aux limites de l’exercice. Nous pouvons nous contorsionner pour ajuster ajuster ou renforcer, ici ou là, les prérogatives des agents de la Suge et du GPSR, mais nous nous heurterons toujours au fait que les gares sont, en l’état du droit, des lieux publics. Cela limite considérablement, sur le plan juridique, nos possibilités d’agir. Je nous invite à poursuivre le travail amorcé, avec raison, par Philippe Tabarot, en menant une réflexion sur le statut de ces lieux, qui pourraient, comme cela a été fait en Espagne, devenir des lieux privés et sécurisés en conséquence. sécurisés en conséquence. Face à l’insécurité dans les transports, le Sénat a toujours fait preuve de responsabilité. C’est, je crois, ce même esprit qui doit aujourd’hui nous guider et nous amener, collectivement, à approuver ce texte. Doter les acteurs du continuum de sécurité de nouveaux moyens

Savary lui même dressait en mars 2020, dans, un bilan mitigé, compte tenu des difficultés rencontrées pour faire appliquer son article relatif à la fiabilisation de l’identité des fraudeurs.

Parallèlement, ainsi que le relève la SNCF sur son réseau, on observe une croissance exponentielle des cas de transport d’objets dangereux : 1 342 personnes ont été signalées pour port et transport illégal d’armes. Les auditions de Jean Castex et de Jean Pierre Farandou, PDG respectivement de la RATP et de la SNCF, ont été à cet égard particulièrement instructives. Selon eux, « l’utilité de cette loi ne fait aucun doute La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, au nom de laquelle je m’exprime devant vous aujourd’hui, a émis un avis favorable sur l’adoption de cette proposition de loi, sous réserve de l’adoption des amendements de son rapporteur pour avis. Nos débats en commission ont été particulièrement riches. À l’aune de ces échanges, il me semble que nous devons garder une chose en tête : la plus grande des restrictions de liberté, c’est lorsque nos concitoyens renoncent à utiliser les transports en commun à certaines plages horaires ou sur certaines lignes. Comme l’a souligné Philippe Tabarot, en Île de France, plus d’une femme sur deux – précisément 51,5 % – redoute d’être agressée ou volée dans les transports en commun. Laisser s’installer l’idée que les transports en commun figurent en tête des espaces les plus criminogènes, c’est renoncer aux évolutions nécessaires pour améliorer l’attractivité des transports collectifs et pour accentuer le report modal vers le système de transport le plus décarboné.

Il est nécessaire d’adapter nos moyens juridiques de répression, qui ne sont plus adaptés aux évolutions des modes opératoires des contrevenants. Ce texte, inspiré par ces situations très concrètes et quotidiennes, a été élaboré en lien étroit avec les acteurs de terrain. Il apporte les évolutions strictement nécessaires à la sécurisation de nos réseaux de transport selon trois volets prioritaires.

attaques. Elle va également au delà des jeux Olympiques et Paralympiques. En définitive, ainsi que l’a résumé Jean Pierre Farandou lors de son audition, cette proposition de loi contribue à apporter un « supplément d’efficacité dans l’action

je salue l’initiative de cette proposition de loi, dont je remercie l’auteur, Philippe Tabarot. L’objectif est de renforcer la sécurité des usagers et des personnels des transports publics face aux incivilités, aux actes de malveillance et aux menaces terroristes. L’actualité vient malheureusement nous rappeler que ces dispositions sont nécessaires pour permettre à nos concitoyens de voyager en sécurité dans nos transports publics. C’est l’une des conditions pour accentuer le report modal vers les transports publics décarbonés, raison pour laquelle le Gouvernement est très attentif Le récent attentat survenu à la gare de Lyon nous rappelle, si besoin était, que nos trains et nos gares ne sont pas à l’abri des tentatives les plus désespérées et les plus violentes. Il nous invite à rechercher en permanence les mesures juridiques et opérationnelles garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux personnels des entreprises publiques de transport, notamment en ce qui concerne les moyens des agents des services de sécurité internes de nos opérateurs de transport, SNCF et RATP, afin de leur permettre d’intervenir le plus rapidement possible, en étroite coopération avec les forces de l’ordre

Les décisions prises ces dernières années pour améliorer la sécurité dans les transports ne sont sans doute pas étrangères à cette amélioration de la tendance. Cela doit nous conduire à poursuivre ce travail de consolidation de notre dispositif de sûreté. Cette proposition de loi s’inscrit ainsi dans la continuité des mesures déjà prises par les gouvernements depuis 2017, notamment au travers de la loi d’orientation des mobilités, de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés de 2021 ou encore de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je rappellerai, pour mémoire, quelques mesures emblématiques, concrètes et efficaces : la généralisation des arrêts à la demande pour les bus nocturnes, l’obligation d’étiquetage des bagages présents à bord des cars express, l’expérimentation du port de caméras individuelles par les agents assermentés des entreprises de transport la possibilité pour les agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP de visionner des images de vidéoprotection transmises en temps réel lorsque lorsqu’ils sont affectés au centre de commandement de la préfecture de police. proposition de loi a le mérite de rappeler de manière très claire les grands enjeux de la sûreté dans les transports publics. Son architecture générale permet de rendre intelligibles les différentes mesures proposées, dans le souci d’être au plus proche du besoin opérationnel. Elle vise ainsi à accroître les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs, à renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation des transports, à utiliser les nouvelles technologies, notamment en matière de vidéoprotection – le Gouvernement souhaitera d’ailleurs introduire une mesure en matière de cybersécurité pour le Grand Paris Express –, à introduire de nouveaux dispositifs pénaux pour réprimer les délits relatifs aux transports et à accentuer le dispositif antifraude. Le Gouvernement tient à saluer le travail réalisé en commission, qui a permis d’enrichir le texte et d’améliorer la rédaction de certains articles. Cette proposition de loi a toute son importance pour améliorer la sécurité de nos concitoyens, qui utilisent chaque jour les transports publics pour leur travail ou leurs loisirs. Elle est d’autant plus nécessaire que nous allons accueillir, dans quelques mois, les jeux Olympiques et Paralympiques à Paris – un événement exceptionnel qui nécessite une mobilisation et une coordination sans précédent de tous les acteurs qui concourent à la sécurité de chacune et de chacun. Certaines dispositions de ce texte visent directement à nous aider à faire face aux enjeux propres à l’organisation d’un tel événement. Je pense notamment à la possibilité donnée à de nouvelles catégories d’agents d’Île de France Mobilités

nos concitoyens sont toujours plus nombreux à emprunter les transports en commun. Ils participent ainsi activement à la lutte contre le dérèglement climatique. Toutefois, les retards et les capacités insuffisantes, notamment dans les transports du quotidien, freinent encore cette dynamique ; il nous appartient de la soutenir. Nos collectivités, en lien avec l’État, travaillent à rendre les Français plus mobiles. Le développement de ces transports ne dépend pas seulement de la construction de nouvelles infrastructures ou de l’offre. En effet, près de la moitié de nos concitoyens disent ne pas se sentir en sécurité dans les transports. Nous ne pouvons et ne devons pas nous satisfaire de cette jeux Olympiques et Paralympiques constitue une formidable opportunité pour notre pays. Ces Jeux seront également une véritable épreuve, tant pour nos opérateurs de transport que pour nos services de sécurité. Nous devons leur donner les moyens de relever le défi. Plus de 15 millions de touristes sont attendus dans la capitale à cette occasion. Outre l’enjeu logistique qu’il représente, cet événement médiatique renforce le risque d’attaque terroriste qui reste, hélas, omniprésent dans notre pays. Beaucoup a déjà été fait ces dernières années pour renforcer la sécurité, mais c’est loin d’être suffisant. Le présent texte vise à aggraver les peines applicables aux infractions commises dans les transports. Il est le fruit de l’excellent travail de son auteur, notre collègue Philippe Tabarot. Ses propositions sont précises et correspondent aux attentes du terrain – croyez moi, j’en sais quelque chose ! Nous considérons que ce message de fermeté est essentiel. Nous ne devons pas accepter que les transports publics soient dégradés par les actes de quelques uns. Les auteurs de fraudes et d’incivilités doivent être sanctionnés rapidement et efficacement. Les usagers doivent pouvoir constater que les règles sont les mêmes pour tous. Ce n’est pas le cas actuellement, alors que le sentiment d’impunité peut parfois régner. Le texte renforce les peines à l’encontre de ceux qui troublent régulièrement la tranquillité des voyageurs. Ces actes, comme le fait de fumer, d’être en état d’ivresse ou encore de tirer sans motif légitime le signal d’alarme, constituent déjà des infractions. Les récidivistes doivent être plus Les récidivistes doivent être plus sévèrement punis. C’est ce que prévoit le texte, tout comme certains amendements que nous aurons le plaisir de vous soumettre. À cet égard, je tiens à souligner la création de la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports Ce nouveau dispositif nous semble pertinent pour sécuriser les transports. Il nous apparaît particulièrement adapté et nécessaire pour lutter plus efficacement contre les agressions sexuelles.

Le texte aborde également la question des difficultés posées par les bagages ou les effets personnels des voyageurs. La disposition visant à pénaliser plus sévèrement l’oubli de bagages dans les transports est lourde, mais il est vrai que celui ci provoque des troubles coûteux et importants pour nos réseaux de transport.

cas d’abandon volontaire de bagages ou de matériaux qui entravent la circulation des trains. Il faut punir sévèrement ces actes qui ne sont rien d’autre que du sabotage. Les transports en commun sont l’un des meilleurs moyens de lutter contre le dérèglement climatique. Ils sont également essentiels au développement de nos territoires et au dynamisme économique de notre pays. Il nous revient de les rendre plus sûrs et de recréer des espaces qui correspondent aux besoins de déplacement de nos concitoyens.

face à la multiplication des actes violents et des incivilités quotidiennes dans les transports en commun et, de façon plus large, dans notre société, faut il faire preuve d’angélisme en pensant que ce phénomène va baisser naturellement ou faut il ajuster le cadre juridique actuel qui régit la sécurité dans les transports publics, afin de réprimer l’ensemble des comportements qui remettent en cause la sécurité et le bien être des usagers ?

C’est dans l’encadrement des mesures de sécurité que se situe la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Nous pouvons compter sur le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’État, qui veillent au respect de nos libertés, comme le démontre la jurisprudence de ces deux institutions – d’ailleurs, respecter leurs décisions devrait aller de soi.

À chaque fois, il leur répondait de regarder si les textes existants ne permettaient pas déjà d’obtenir les résultats recherchés. Je ne doute pas que notre collègue Philippe Tabarot ait entrepris cette démarche avant de déposer la présente proposition de loi, le 28 décembre dernier.

Il ne bouleverse pas donc un ordre juridique établi ; il s’inscrit plutôt dans la continuité. En dix neuf articles, le texte de notre collègue, soutenu par nombre d’entre nous, vise à répondre tant à différentes lacunes de la loi en matière de sécurité dans les transports qu’à de nouvelles formes de délinquance et d’incivisme. Ainsi, combien de fois par jour les lignes de métro parisiennes sont elles bloquées par des oublis de bagages ? Voilà quelques années, ce phénomène était rarissime. Aujourd’hui, il est quotidien, qu’il résulte d’actes intentionnels ou non.

Pour relativiser les conséquences des évolutions soumises à notre approbation, je me permets de vous rappeler qu’en Chine l’accès aux transports en commun se fait la reconnaissance faciale. Ce système a été mis en place prétendument afin de fluidifier les entrées dans les transports. En réalité, il s’agit bien entendu de contrôler les déplacements des usagers et non de penser à leur bien être ou à leur sécurité physique. Je n’entrerai pas dans la bataille des chiffres sur la hausse ou la baisse de la délinquance dans les transports en commun. Il faut être réaliste : celle ci progresse tant en raison de l’augmentation

Ce transfert, cette délégation de compétences, ce que vous appelez le « continuum de sécurité », devient trop souvent un « continuum sécuritaire ». Mon collègue Thomas Dossus avait déjà défendu cette position lors de l’examen de la loi Sécurité globale. Il avait alerté sur cette tendance à la confusion des genres.

Certes, les attaques récentes que notre pays a connues doivent nous faire réfléchir à de possibles améliorations du cadre législatif. L’organisation prochaine de grands événements comme les jeux Olympiques alimente le questionnement sur les enjeux de sécurité de notre pays.

de loi a été largement modifiée par les travaux des rapporteurs, qui ont tenté, à juste titre, de limiter les risques de censure en procédant à un toilettage juridique des mesures les plus problématiques.

mais le pragmatisme, c’est mettre les moyens là où ils sont utiles. Le pragmatisme ne doit pas se faire au prix d’une course vers la société de surveillance, de l’emploi de technologies d’enregistrement sans contrôle, de la multiplication des fichiers, Je m’attarderai sur la question des fouilles et des palpations, ainsi que sur celle des saisies. Notre commission, dans sa grande sagesse, a su rectifier le tir concernant l’article 1 sur les saisies, dont le dispositif était juridiquement bien trop bancal. Désormais, les autorisations de palpations sont placées sous le régime d’autorisation du préfet, ce qui est déjà mieux, mais pas tout à fait satisfaisant

Que dire aussi de l’article 12 et de son catalogue à la Prévert de nouvelles incriminations allant du transport d’une arme à feu à la détention d’un mauvais titre de transport, en passant par le fait de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou des tapages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, sans parler de l’alinéa criminalisant la mendicité Un ronfleur, un passager ayant un clavier trop bruyant et une personne transportant une arme à feu risqueront désormais les mêmes peines : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende – moi qui oublie souvent ma casquette… Nous voyons bien l’absurdité de cet article que nous tenterons de modifier. Au delà, nous n’avons pas été convaincus sur la question de la perception de l’intentionnalité dans ces incriminations. Qu’est ce qui sera considéré comme intentionnel ? Selon quels critères objectifs ? Le risque d’arbitraire nous paraît bien trop important.

sur l’utilisation des algorithmes ou des caméras et sur bien d’autres aspects problématiques de ce texte. Mes chers collègues, les gares ferroviaires, les stations de métro et de bus, les réseaux ferrés ainsi que les véhicules de transport sont, par nature, comme le rappelait la rapporteure, vulnérables à différentes menaces existantes et identifiées.

Il s’agit de la troisième en quelques années, après la loi Savary de 2016 et la loi dite Sécurité globale de 2021. Je regrette le choix de ce véhicule législatif, qui ne nous permet d’appuyer nos débats ni sur une étude d’impact ni sur un avis du Conseil d’État. Ce n’est pas un détail tant les multiples dispositions de ce texte risquent de bouleverser le quotidien de millions d’usagers des transports en commun et du rail. Nous débattons dans un contexte sécuritaire tendu, quelques jours après l’attaque au couteau en gare de Lyon, qui a fait – malheureusement – plusieurs blessés.

cette réalité ne peut pas tout justifier. Je regrette que ce texte soit moins une proposition de loi qu’un catalogue de mesures à objectifs distincts : prévention du risque terroriste, lutte contre les incivilités ou encore contre la fraude. On passe d’un article à l’autre sans cohérence globale. Ces sujets auraient pourtant mérité davantage de considération. De plus, sous couvert d’efficacité, cette proposition de loi acte une nouvelle fois le désengagement de l’État du domaine de la sécurité, un secteur pourtant régalien par excellence. Désormais, sur décision du préfet de police, les agents de la Suge ou du GPSR pourront réaliser des palpations préventives de sécurité et se verront attribuer un droit de poursuite des contrevenants. Les agents de sécurité privée ne sont pas des policiers ou des gendarmes. De quelles formations bénéficieront ils pour appréhender ces nouvelles missions ? Sur quelles données objectives un préfet prendra t il la décision d’autoriser ces mesures de palpation préventive ? De plus, comme l’avait si bien dit notre ancienne collègue Éliane Assassi lors du débat sur la loi Savary : « Cette proposition de loi oublie la spécificité de la mission de sûreté, […] à savoir la sécurité des infrastructures et la nécessité d’assurer la fluidité et la continuité de la circulation. Ces mots n’ont pas perdu leur actualité ; or, sur ce point, votre texte reste muet. Vous proposez aussi que le renforcement du continuum de sécurité repose sur les agents des polices municipales, qui seraient désormais autorisés par convention à accéder aux véhicules et aux espaces de transport. au détour d’un texte, voilà une drôle de prérogative nouvelle pour nos communes ! Avez vous bien conscience, mes chers collègues, que nos polices municipales sont diverses et territorialisées ? Comment sera appliqué le pouvoir de police du maire dans les transports en commun ? À moins que vous ne partiez déjà du principe que les trains resteront en gare – les usagers retenus à quai apprécieront… Je suis également inquiet de constater que ce texte autorise, sous couvert de placer la technologie au service de la sûreté dans les transports, le recours à un traitement algorithmique des images issues des systèmes de vidéoprotection ainsi que la captation du son dans les véhicules. Cela participe d’un mouvement vers une forme de sécurité prédictive, fondée sur les seuls indicateurs de risques. Il est connu que ces dispositifs présentent des limites et des biais discutables. Il en va de même pour le fichage des auteurs d’infraction dans les transports, retoqué par le Conseil d’État en 2016, mais réintroduit ici sous une nouvelle rédaction. De plus, votre texte ne fait que durcir les sanctions applicables à des délits déjà sanctionnés par la loi. Je m’interroge aussi sur votre vision du service public. Depuis plusieurs années, les politiques de réduction du personnel ont limité la présence en gare : la plupart des guichets sont fermés, quand ce ne sont pas les gares elles mêmes… Et que dire des conditions de transport, qui se sont largement dégradées.

ou les parents avec leurs poussettes ? Cette situation crée un climat de tension propice à exacerber le sentiment d’insécurité. La priorité est donc de réintroduire de l’humain dans nos gares et nos trains, au service du public, dans une approche positive et accueillante, et d’investir pour nos transports afin de les rendre eux aussi positifs et accueillants. Nous sommes tous persuadés que la sécurité et la tranquillité publiques dans les transports sont des sujets de société sensibles et importants. Ils sont aussi le gage de la transition nécessaire vers des modes de transport décarbonés. Il nous faut donc prendre le temps de débattre largement et avec sérieux et éviter de créer des spécificités sécuritaires d’un espace public à l’autre. Pour toutes ces raisons, le groupe CRCE K votera contre ce texte.

Cet événement, malheureusement loin d’être inédit, ravive le sujet de préoccupation constant qu’est l’insécurité dans les transports, enjeu d’autant plus important à l’approche des jeux Olympiques et Paralympiques. En sus de la menace terroriste, qui reste à un niveau élevé, 111 531 personnes ont été victimes de vols et violences dans les transports en commun en 2023, dont 62 % en Île de France. Une réalité qui a poussé la RATP à mettre en place l’arrêt à la demande dans les bus de son réseau, après vingt deux Et une réalité d’autant plus forte pour les femmes : 87 % d’entre elles déclarent avoir été victimes de violences sexuelles et sexistes dans les transports. Cette proposition de loi part de ce constat de vulnérabilité et du manque d’efficacité du cadre juridique de répression aujourd’hui en place. objectif est d’octroyer aux agents les moyens nécessaires à la sécurisation des transports en commun et de combler les lacunes de la législation pénale en vigueur. Le groupe RDSE souscrit à cette ambition. Pour faciliter leur mobilité, d’abord, il est proposé d’élargir le périmètre d’intervention des agents de sécurité des transports aux abords immédiats des gares, si l’infraction a été commise dans la gare et si le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie. Une mesure de bon sens, tout comme celle leur permettant d’intervenir dans les réseaux de transport urbains connectés aux gares. Nous souscrivons aussi à la possibilité offerte aux maires et présidents d’EPCI de conclure une convention avec un exploitant de service de transport public afin de permettre l’accès libre des policiers municipaux et des gardes champêtres aux gares et aux trains en circulation sur leur territoire. Toutes ces mesures permettront de renforcer le continuum de sécurité. La création d’une interdiction d’entrée en gare nous apparaît également opportune pour les personnes troublant l’ordre public, compromettant la sécurité ou refusant de se soumettre à des palpations de sécurité. Nous espérons toutefois qu’une forme de retenue sera appliquée concernant la fouille des bagages. De la même manière, bien qu’il s’agisse d’une infraction rarement sanctionnée, une amende de 7 500 euros pour mendicité, même répétée, nous semble au mieux inapplicable. dresse la liste d’un grand nombre d’incivilités ouvrant la porte à une sanction pour délit d’habitude. Si ces espaces publics nécessitent des comportements adaptés, priorité doit être donnée au traitement des comportements dangereux. le recours aux caméras piétons, nous aurions préféré attendre le bilan de l’expérience qui est en cours avant toute pérennisation. Nous saluons toutefois la mise en place de l’expérimentation permettant aux chauffeurs de bus et de car d’utiliser un tel dispositif. dispositif. Le drame survenu à Bayonne en 2020, avec la mort d’un conducteur, nous rappelle que les chauffeurs sont en première ligne face à des usagers de plus en plus violents. Le nombre d’agressions sur le personnel ayant donné lieu à un arrêt de travail était ainsi en hausse de 14 % en 2022. Ces outils permettent de dissuader, de capter les situations à risque et d’avertir les services de sécurité en cas de danger imminent. Je tiens à rappeler ici que le groupe RDSE est attaché à préserver l’équilibre entre sécurité et libertés publiques, mais qu’il regarde le sujet avec beaucoup de pragmatisme. D’autres mesures, qui risquaient de remettre en cause certaines libertés individuelles, ont été modifiées ou supprimées en commission. Nous soutenons ainsi le travail d’équilibre de la rapporteure, qui a proposé la suppression de plusieurs mesures que nous jugions excessives : la saisie d’objets licites sans caractère de dangerosité ; la collecte et le traitement de données sensibles par les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP ; ou encore la captation sonore dans les transports. Enfin, nous proposerons un amendement visant à supprimer l’amende de 2 500 euros à l’encontre des voyageurs oubliant leur valise, qui nous paraît disproportionnée. Je pense, par exemple, à la mère de famille chargée de ses enfants et de ses bagages, qui descend du train en oubliant l’un d’eux – je parle des bagages et non, bien sûr, des enfants ! Elle ne peut décemment pas être sanctionnée pour cette inattention, bien que fâcheuse.

les transports collectifs concernent chaque jour plusieurs millions de nos compatriotes. Le développement, l’accessibilité et la sécurité des transports en commun sont au cœur des enjeux visant à faire de ces derniers des leviers pour la transition écologique et énergétique.

Les agents de sûreté des transports en commun ont des responsabilités importantes pour la protection des usagers. Aux côtés des forces de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les polices spéciales de la Suge et du GPSR sont des vigies opérationnelles œuvrant à notre sûreté. Gardons aussi à l’esprit que notre pays est une destination touristique reconnue. Or une grande majorité des visiteurs, en tout cas en région parisienne, sont amenés à emprunter les transports collectifs. de loi déposée par notre collègue Philippe Tabarot a le mérite d’ouvrir le débat sur les améliorations à apporter afin de mieux répondre aux défis contemporains et à venir. La persistance des violences sexistes et sexuelles, des vols, des fraudes et de la menace terroriste vient en effet alourdir un climat déjà dégradé. Le statut particulier de la SNCF et de la RATP a conduit le législateur à leur accorder des prérogatives spécifiques, consacrées par la loi du 12 juillet 1983.

Ce travail était nécessaire tant – il faut bien le dire – la rédaction initiale pouvait susciter quelques réserves, notamment sur les processus de captation des sons dans les véhicules ferroviaires. Le travail mené par Mme la rapporteure a également permis d’enrichir et de compléter la proposition de loi. Nous tenons sincèrement à saluer son travail. Ce texte, résolument tourné vers le renforcement du continuum de sécurité et l’approfondissement de notre arsenal pénal, apporte sur certains points des avancées extrêmement pertinentes. L’usage à titre expérimental d’une caméra piéton par les conducteurs de bus est une bonne mesure. Ces agents ne sont pas seulement la cible de comportements vexatoires ou intimidants, mais parfois l’objet d’une violence non contenue et revendiquée.

La pérennisation de ce dispositif pour les agents de contrôle des transports concourt utilement à promouvoir la sûreté. Nous saluons également les prérogatives supplémentaires qui seraient attribuées aux agents de contrôle et de sûreté, en particulier la création d’un droit de communication de données fiscales en vue de fiabiliser encore le recouvrement des amendes.

s’il n’est pas négligeable de mieux appréhender et de faire reculer le phénomène des oublis de bagages, qui entrave la circulation sur les réseaux, en faire un délit ne nous paraît pas la solution législative la plus évidente ni la solution opérationnelle la plus adaptée. L’extension du périmètre d’intervention des agents de la Suge et du GPSR en dehors des emprises et véhicules de transport part d’une intention louable, celle de desserrer un étau parfois trop restrictif. Toutefois, jusqu’où cette extension est elle fixée ? La difficulté est qu’un élargissement géographique imprécis ou trop vaste viendrait fragiliser les équilibres et altérer la répartition des pouvoirs entre police spéciale, d’une part, et police générale, d’autre part. Nous avons eu des débats en commission sur ce sujet. devons répondre est bien celle de l’amélioration des moyens juridiques et opérationnels en direction de ceux qui nous protègent chaque jour et dans la durée. Nos intentions ne suffisent pas ; il nous faut aussi assurer l’opérationnalité des mesures que nous votons. de cette proposition de loi, il nous est proposé de mieux accompagner les forces de sécurité. C’est une intention que nous saluons et que nous soutenons, mais nous sommes arrivés au bout de ce que nous pouvions faire sans un vrai travail de refonte du droit existant. Encore une fois, cette proposition de loi apporte un certain nombre de changements, par petites touches, mais il faudra une réflexion beaucoup plus profonde et globale si l’on veut véritablement répondre aux besoins des forces de sécurité et à ceux des usagers.

les utilisateurs des systèmes de transport. La loi Savary Leroux et la loi Sécurité globale de 2021 sont venues renforcer le dispositif en allant plus loin à chaque fois, en octroyant de nouvelles prérogatives aux acteurs de la sécurité et en articulant au mieux les attributions de chacun.

La proposition de loi de notre collègue, largement amendée par la commission des lois, vise à aller encore beaucoup plus loin et à attribuer des prérogatives supplémentaires, en renforçant notamment le continuum de sécurité et en étendant la surveillance par le recours à de nouvelles technologies.

article 8 permet la mise en place d’un numéro téléphonique unique, ce qui nous paraît aller dans le bon sens. Enfin, il faut donner des outils aux sociétés de transport pour lutter contre les personnes malveillantes qui ne respectent pas les règles – là aussi, nous sommes d’accord.

On pourrait multiplier les chiffres, mais je n’en retiendrai qu’un : à elle seule, l’Île de France représente deux tiers des victimes des vols et violences dans les transports en commun. Je suis une femme et comme toutes les femmes je revendique l’égalité du droit à emprunter les transports en commun en toute sécurité pour le travail, la vie quotidienne, les loisirs, tôt le matin et jusque tard le soir. Je comprends le sentiment d’insécurité et parfois la terreur de tant de femmes, en particulier parmi les plus modestes, qui empruntent les transports en commun à des heures très matinales ou très tardives, non pas, à titre principal, parce qu’elles souhaitent contribuer à l’indispensable décarbonation des transports, mais parce qu’elles n’ont tout simplement pas d’autre choix. Beaucoup de femmes hésitent d’ailleurs à les emprunter. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à utiliser les transports vers Paris. Elles sont moins nombreuses que les hommes à utiliser les transports dans les zones sensibles. Plus la fin de journée avance, moins les femmes y sont présentes : leur proportion diminue de moitié. Et les femmes ont raison d’avoir peur : elles représentent 60 % des victimes de violences. Enfin, je suis une mère et je partage la colère de tant de mères, parisiennes ou franciliennes, dont l’enfant ou l’adolescent a été suivi, agressé ou racketté dans le métro ou à ses abords.

des bandes agressives, qui font tant de mal et restent si souvent impunis. Si la situation est aussi grave, ce n’est pas faute d’actions, et même d’actions très vigoureuses, de la part de Valérie Pécresse, de la région Île de France, d’IDFM,

Pour faire face à cette montée inquiétante de la violence et à la diversification toujours plus grande des modes opératoires, pour restaurer la confiance, il faut donner aux opérateurs tous les moyens juridiques de s’adapter et d’aller plus loin.

Les policiers municipaux pourront circuler et intervenir dans les gares et les trains. Le texte permettra également de faciliter le recours aux caméras piétons : ce sera très utile pour la sécurité des agents comme pour le traitement des dossiers. Enfin, Enfin, il est bien entendu nécessaire d’adapter la réponse pénale. La création d’un délit d’incivilité d’habitude est très attendue par les acteurs du secteur, mais plus largement par tous ceux qui trouvent insupportables ces comportements nuisibles et non sanctionnés qui pourrissent la vie de tous au quotidien.

Non, nous ne pouvons conditionner des palpations de sécurité dans les transports aux seuls cas où le préfet de police aurait pris, en amont, un arrêté spécifique, parce qu’il y a une manifestation ou une menace à l’ordre public sur un certain périmètre. Il est des situations d’urgence, avec un risque immédiat pour la sécurité des personnes, où il faut intervenir et où seuls les agents de la sûreté des transports sont à même de le faire. Nous ne pouvons non plus priver les agents de sécurité d’écouter ce qui se passe dans une rame ou un bus, alors que la sécurité des personnes est immédiatement menacée par un accident ou par des personnes violentes

Certains objets, qui ne sont pas des armes, peuvent en certaines circonstances se révéler dangereux pour les autres voyageurs. Ils ne sauraient donc avoir leur place dans les transports publics. La sécurité desdits transports est essentielle à la qualité de vie des Français, comme à celle des millions de touristes que nous accueillons chaque année – et je ne pense pas seulement à cette année olympique. C’est pourquoi nous devons vraiment aller aussi loin que possible. Pour les agents de sécurité, rien n’est pire que l’impuissance. Pour les voyageurs, rien n’est pire que le sentiment d’insécurité permanent, rien n’est pire que des agressions, de surcroît impunies faute de moyens juridiques idoines. Il n’y a pas de liberté d’aller et venir sans transports sûrs. Pour l’ensemble de ces raisons, je voterai ce texte, amendé. Bravo ! La parole

les gares, les métros sont des lieux où des milliers de personnes se croisent chaque jour, chacune avec son propre itinéraire, ses propres préoccupations. Pourtant, au milieu de cette diversité, il y a une constante : l’insécurité, la peur de devenir la cible d’agresseurs, la peur de se retrouver pris dans une bagarre, la peur de ne pas rentrer chez soi sain et sauf pour un simple regard. La violence dans les transports en commun revêt de nombreuses formes. Il y a bien sûr les agressions physiques, ces actes lâches qui laissent des cicatrices sur les victimes, mais il y a aussi la violence verbale, les insultes, les propos racistes, sexistes ou homophobes, qui empoisonnent l’atmosphère et augmentent l’insécurité. Et n’oublions pas la violence psychologique, cette pression constante qui pèse sur les voyageurs, qui regardent par dessus leur épaule à chaque bruit suspect, se demandant si ce sera leur arrêt ou celui de l’agresseur. Certains diront que la violence dans les transports en commun est un phénomène de société inévitable, mais ce n’est pas vrai. Nous ne devrions jamais accepter la violence comme une norme sociale. Nous avons le droit de nous déplacer en toute sécurité, sans craindre pour notre intégrité physique. En 2019, 13 % des vols dans les transports en commun se sont finis par des actes violents. En 2022,

le sujet. La violence dans les transports en commun est un problème urgent, qui nécessite une réponse collective. En refusant de rester silencieux, en demandant des comptes aux autorités, nous pouvons faire de nos bus et de nos rames des espaces sûrs et accueillants pour tous. Ne restons pas les témoins passifs de cette injustice : il faut agir. Nous soutiendrons bien évidemment cette proposition de loi. La parole

chers collègues, ce texte est intéressant. Comme d’autres avant moi, je veux remercier chaleureusement Philippe Tabarot, qui est bien souvent mon complice dans les affaires ferroviaires, mais qui ne le sera peut être pas aujourd’hui…

aveuglé par une idéologie d’un autre temps. Loin de nous l’idée de minimiser les questions de sécurité et d’incivilité dans les transports collectifs. Je suis et nous en sommes des usagers fréquents, même quotidiens pour nombre d’entre nous. Et parce que le groupe socialiste ne les minimise pas, je veux concentrer mon propos sur le travail des agents dont la mission est justement de protéger et d’assurer la tranquillité des usagers.

Si je comprends et puis partager un certain nombre des intentions de Philippe Tabarot, je ne voudrais pas que ce texte apporte plus de questions que de réponses. Prenons garde à ne pas déshabiller les uns pour habiller les autres. La Suge et le GPSR ont fait depuis des années la preuve de leur pertinence et de leur efficacité. Attention à ne pas ouvrir sans condition les capacités d’intervention des polices municipales, par exemple, dans ces nouveaux espaces. Dans la même veine, nous devons éviter de trop faciliter la compensation du manque d’effectifs de la Suge et du GPSR par l’extension des possibilités de recours à des agents privés,

Ayons garde de ne pas introduire du mal être parmi les agents de nos entreprises publiques, surtout à quelques semaines des jeux Olympiques et Paralympiques et à l’heure de l’ouverture à la concurrence des réseaux franciliens et ferroviaires partout en France. Après

des effectifs de contrôle et de lutte antifraude entre différents lots, et donc potentiellement différents opérateurs, rendra par définition plus difficile la constitution de brigades

Alors que les jeux Olympiques et Paralympiques approchent, nous avons besoin d’un cadre approprié pour la sécurité de nos transports publics, à Paris et sur tout le territoire. Nos transports publics prennent en charge 10 millions de voyageurs chaque jour.

Limiter le nombre d’actes de malveillance dans les transports en commun est devenu un enjeu crucial. Nos gares, nos stations et nos rames restent des lieux attractifs qui favorisent différentes violences, incivilités et menaces. La sécurité reste une exigence primordiale, mais il est difficile de mobiliser en tout temps et en tout point de nos réseaux une police nationale déjà abondamment sollicitée. Dans certains cas, elle ne peut intervenir qu’en dernier recours. Pour assurer le continuum de sécurité, il faut donc s’appuyer sur celles et ceux qui garantissent la sûreté dans nos transports. Les agents de la Suge ou du GPSR, s’il s’agit de la RATP, disposent d’une connaissance précieuse de ce terrain fluide et mouvant. Ils se heurtent pourtant aux contraintes d’un cadre limité, alors qu’ils sont formés et compétents. Il existe des trous dans la raquette, alors que nous disposons d’agents performants, dont le travail pourrait même soulager

Si les délinquants méprisent la loi, ils en connaissent très bien les insuffisances et les lacunes. Ils ont beau la bafouer, ils savent habilement invoquer la moindre de ses faiblesses dans les prétoires. Ne leur offrons pas un moyen de défense supplémentaire en maintenant une législation incomplète et inadaptée. de la compétence des agents de la Suge et du GPSR pour constater et poursuivre les infractions sur les seules emprises immobilières et véhicules de transport soulève inévitablement le problème du périmètre d’intervention.

N’encourageons pas les délinquants et les criminels avec de bien picrocholines querelles de territoires administratifs. Aussi, pour rester fidèle à la jurisprudence constitutionnelle qui interdit le transfert à des personnes privées des compétences de police générale, la commission des lois a précisé que l’intervention aux abords immédiats est bien un « droit de poursuite

Pour des voyageurs qui n’avaient rien demandé, ce sont parfois des heures gâchées ou des demi journées perdues. Aussi, je me réjouis que soit institué un nouveau délit d’oubli des bagages. Après tout, l’imprudence et la négligence sont bien déjà prises en compte dans notre code pénal et peuvent être sanctionnées.

un texte important et attendu par les opérateurs de transport collectif. Il aidera surtout les usagers, qui ont plus que jamais droit à la sécurité quand ils voyagent et se déplacent.

plus la coopération entre les forces de sécurité intérieure de l’État et les forces de sécurité internes des opérateurs de transport. La discussion

Seul un officier de police judiciaire, policier ou gendarme, a compétence pour effectuer ces gestes dans les cas de flagrant délit, de commission rogatoire ou d’enquête préliminaire. Les agents de transport peuvent seulement inspecter visuellement des bagages à main avec le consentement de la personne. L’exigence de l’article 66 de la Constitution ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui ne sont pas mis à la disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes. Enfin, selon les dispositions de l’article R. 434 16 du code de la sécurité intérieure, la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté et ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité de l’agent qui l’accomplit

Je rappelle que, en l’état du droit, de telles palpations sont systématiquement subordonnées à la prise d’un arrêté préfectoral instituant un périmètre de sécurité ou constatant des circonstances particulières

quelques instants et qui vise justement à rétablir la rédaction de l’article 1 dans sa version initiale, avec deux conséquences. La première est de permettre aux agents de la Suge et du GPSR de procéder à des palpations de sécurité si des éléments laissent à penser qu’une personne pourrait

à réaliser des palpations administratives de sécurité lorsqu’il existe des éléments objectifs laissant à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des voyageurs. Cet article permet à ces mêmes agents de se saisir des objets dangereux susceptibles d’être introduits dans les véhicules de transport. Le danger pouvant survenir de manière inattendue, le fait de subordonner la réalisation de telles palpations à une décision administrative préalable ne répond qu’imparfaitement à la réalité du risque qui menace chaque jour les voyageurs, les personnels et les usagers des gares.

à retirer et remettre aux forces de sécurité intérieure des armes classifiées qu’ils découvrent lors des fouilles, mais ne peuvent saisir d’autres objets dangereux pourtant susceptibles de constituer des armes par destination, tels que couteaux de boucher, pics à glace, cutters, battes de baseball et j’en passe… Lorsqu’un officier de police judiciaire, appelé par les agents de la Suge ou du GPSR, n’est pas en mesure de se déplacer, l’individu est laissé libre avec les objets dangereux en sa possession. Les agents sont autorisés à retirer et remettre aux forces de sécurité intérieure des armes classifiées qu’ils découvrent lors des fouilles, mais ne peuvent saisir d’autres objets dangereux pourtant susceptibles de constituer des armes par destination,

Merci,